La séance est reprise alors nous reprenons la discussion du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur et dans la discussion des articles que nous sommes parvenus à l'amendement numéro 183 au sein du rapport annexé à l'article alors 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 183 il est retiré, madame la présidente, retirer merci madame la présidente, le 142 monsieur dessus. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, on va évoquer un sujet qui vous est cher cher dans tous les sens du terme, puisqu'on va parler vidéo-surveillance et tout le taux long du rapport, il est rappelé que les crédits dédiés au déploiement des caméras de surveillance par les collectivités seront doublés si l'aspect des moyens et donc largement documentée à aucun moment, il est fait mention de l'efficacité au des finalités de ce dispositif, permettez-moi de vous rappeler que la Cour des comptes s'interroge à ce sujet dans son rapport d'octobre 2020, l'institution de la rue Cambon pointent l'absence de lien entre vidéo-surveillance et baisse de la délinquance elle cosigne questionne ainsi des dispositifs au coût très importants et dont l'efficacité reste donc à démontrer une autre tu de récentes menées en Isère, à la demande du Centre de recherche de la gendarmerie nationale, conclut aussi un apport très marginal de la vidéosurveillance dans la résolution d'enquête judiciaire mais aussi. donc le rapport Ce rapport propose quelques pistes pour améliorer mais donc il est quand même temps d'évaluer sérieusement cette politique de vidéosurveillance ce rapport annexé souhaite ouvrir les données de votre ministère et faire la part belle aux recherches académiques, nous vous proposons donc de permettre aux chercheurs qui le souhaitent de s'intéresser à la politique de vidéosurveillance du ministère leur éclairage est de nature à améliorer la décision et l'évaluation de nos politiques publiques, c'est le but de cet amendement. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui on on a eu le débat juste avant l'interruption, le même débat : avis défavorable pour les mêmes raisons. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre, même avis je mets donc aux voix l'amendement 142 qui a reçu, donc un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il n'est donc pas adopté l'amendement 143 messieurs dessus. Merci madame la présidente, le recul de la présence des services publics touche toutes les politiques publiques françaises dans le cas qui nous concerne et cela été justement rappelé dans le rapport que nous étudions les fermetures de commissariats ont été importantes, 500 brigades de gendarmerie fermé en 15 ans, 20 commissariats, fermé depuis 2008 10 arrondissements supprimer 9 jumelée depuis 2014 ce constat devrait tous nous interpeller. Le rapport annexé fait ainsi preuve d'une prise de conscience salutaire et que nous proposons d'enrichir par une simple formule un principe simple : pas de fermeture de commissariat ou de brigades de gendarmerie sans consultation du maire, c'est un principe qui a déjà été mise en place dans les classes dans pour les classes d'enseignement primaire et qui a été chaleureusement accueilli par les élus locaux sont toutefois hélas, aux dernières nouvelles, avoir été pérennisé en effet pour l'école, comme pour la sécurité, les maires connaissent les besoins de leur commune et les problématiques des habitantes et des habitants, ils sont donc à même d'éclairer la politique d'implantation décidée par l'État central, si un maire insiste pour garder un commissariat ouvert c'est qu'il sait que ses moyens en terme de police municipale sont insuffisants pour faire le travail et que la sécurité de ses administrés peut en pâtir le dialogue entre élus locaux et ministère de l'Intérieur, doit être améliorée, c'est ce que nous vous proposons avec cet amendement. Merci l'avis de la commission monsieur le. ça demandé en commission que cet amendement fut rectifier parce que ils soumettaient la décision à un accord préalable du maire, là, il a été rectifiée consultation du maire, le fait que l'on consulte la c'est Lemaire et que dans d'autres cas, c'est le conseil municipal, par exemple pour les fermetures de classes, me semble être une bonne mesure, c'est une consultation et après le l'exécutif décide ce qu'il a décidé donc favorable pour une fois. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre, vous êtes favorable donc, et donc je mets aux voix l'amendement 143 qui a reçu un avis favorable de la commission et du gouvernement qui est pour, qui est contrat qui s'abstient donc adopté 3 amendements identiques. L'amendement vingt-trois Monsieur Durand. Monsieur le ministre, madame la présidente, mes chers collègues, dans de nombreux territoires les territoires ont de de besoins en matière de reconstruction à 9 de leur caserne de gendarmerie ses casernes vétustes ont besoin d'être remplacés dans les prochaines années afin que gendarmes travaillent et soit dans de meilleures conditions, c'est le cas en Meurthe-et-Moselle, dans la Nièvre et dans bien d'autres départements ces casernes situées en milieu rural, ne répondent pas aux normes actuelles de confort et de sécurité, avec un impact donc sur les conditions de travail, la vie des gendarmes et de leurs familles sur l'attractivité également des affectations des gendarmes, le décret de 2016, 2000 16884 relatives aux conditions de réalisation de ces logements dispose que l'état garantit un loyer au maître d'ouvrage d'un montant plafonné est proportionnel au nombre d'unités de logement de la caserne ce loyer, donc qui est versée aux maîtres d'ouvrage et donc décorrélés de la taille des casernes, dont les surfaces comprennent, en plus des logements, les locaux indispensables au service ces locaux nécessaires, le locaux nécessaire, quelle que soit la taille de la caserne représente donc un coût fixe importants qui pénalise les petites casernes, dont le coût de revient l'unitaire par logement devient hein, par conséquent, infinançables est supérieur à la moyenne des grandes caserne dans ces conditions, les auteurs du présent amendement propose au gouvernement de modifier ce décret, le décret de 2013 sur les modalités d'attribution des subventions aux collectivités locales pour la construire une gendarmerie en ajustant la subvention d'investissement collectivités en fonction du nombre d'unités de logement des casernes, par exemple, les casernes de moi de 9 unités de logement recevront une subvention de 30 pourrait être ensuite dégressive, il est proposé également d'ajuster la durée de Dubaï au sel à celui à cette durée, pardon des remboursements des emprunts contractés, c'est ainsi qu'on pourrait traiter de manière équitable, les territoires ruraux et ce besoin de sécurité qui existe aussi en matière de territoire et d'espace rural merci. Merci l'amendement 211 Monsieur Paul. Oui merci madame la présidente, le présent amendement est identique à l'amendement suivant de la commission des lois, avec laquelle nous partageons une même préoccupation en effet la création de 200 nouvelles brigades constitue certes une bonne mesure pour permettre à la gendarmerie de se rapprocher, de se rapprocher des territoires en revanche créer une brigade sur le papier, une chose construire les locaux professionnels et les logements pour l'accueillir en est une autre d'abord ce n'est pas la même échelle de temps, ensuite il faut des moyens d'investissement car il n'existe toujours pas de locaux vacants qu'ils qu'ils à parlé de collectivités territoriale ou à l'État, monsieur le Ministre, ces moyens sont souvent fournis par les collectivités locales à travers divers dispositifs juridiques malgré certaines aides prévues par les textes, ce n'est pas neutre financièrement pour lesquels collectivités les dépenses d'investissement sont comptabilisés dans les Budgets locaux il existe donc un risque d'inégalité des collectivités devant ses dépenses à effectuer notre amendement vise ainsi à permet de l'adaptation des règles budgétaires et comptables, ainsi qu'un meilleur soutien financier afin que seuls des critères liés à la délinquance et au besoin de sécurité publique soient pris en compte pour l'installation de cette nouvelle brigade

et qui recouvre exactement ce que les collègues ont ont évoqué de manière très précise : Monsieur le Ministre, Kant, vous allez décider de la construction de 200 nouvelle caserne de gendarmerie ou quand, dans les territoires des casernes vont être agrandi pour les besoins nécessaires des gendarmes et de leur famille, les investissements vont être portés par les collectivités, le territoriales, commune, intercommunalité et parfois vous, on va avoir recours à des syndicats départementaux à des bailleurs sociaux qui vont porter l'immobilier de ces constructions pour la durée de l'utilisation de ces casernes par l'État par la gendarmerie ces casernes vont être construites, elles vont représenter une charge financière qui, qui n'est pas négligeable notamment à le ça va, ça va continuer de la dette pour ces collectivités, ça va constituer des dépenses de fonctionnement compensés très souvent fort heureusement par des par une recette de fonctionnement équivalentes, mais cette dette ses dépenses et ses recettes de fonctionnement peuvent être de nature à déstructurer les ratios financiers des collectivités en question, on est dans une période dans laquelle évidemment le, le fait de pouvoir emprunter sur les marchés est un enjeu, le fait de ne pas être surendettés en tant collectivité est un enjeu et je crois que dans tous nos départements, on a été les uns et les autres, alerté par ces situations-là, l'amendement en question est un un moment dans le rapport, qui vise à vous sensibiliser sur cette question là et à essayer de trouver, j'imagine avec Bercy, des solutions qui permettront de manière intelligente de si possible des en tout cas de traiter à part cette dette et ses dépenses et recettes de fonctionnement pour que les ratios budgétaires de nos collectivités ne soit pas trop affecté, je vous remercie. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Bien, madame la présidente, je voudrais donner un avis favorable aux au moment des du rapporteur et donc des des 2 intervenants, quelles que soient les les groupes politiques, je sais pas si Monsieur Snyder Jacques hein, c'est une bonne chose que de modifier le décret comme vous l'entendez, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sujet

Je pense que il faut aussi que l'infection à c'est quoi une caserne de gendarmerie de demain, est ce que les militaires voudront toujours vivre avec leur famille dans ses casernes. C'est pas une guerre question facile à répondre, parce que ça tient la de la gendarmerie, mais ça tient aussi aux nouvelle composition familiale du fonctionnement de la vie de nos concitoyens militaire qui choisit de gendarmerie parfois pour garder les familles dans des territoires, il vaut mieux peut-être selon les territoires qui vivent dans un habitat. Je lui dis fuck à la caserne, en tout cas la question peut se poser, je n'ai pas apporté de réponse mais je sais qu'avec les élections générales, la gendarmerie, nous y réfléchissons, la 2ème question qu'évoque notamment le le rapporteur Hervé c'est quel est le modèle financier qui permet à bien sûr à la collectivité, de participer, ça me paraît pas délirant que le faire et d'ailleurs, dans certains cas, vous savez bien qu'il y a aussi un retour son enrichissement qui était intéressant pour certaines communes, mais pour à peu près 40 % des autres cas, les collectivités locales ont été emmenés soit dans des dépenses qui était trop importante pour même quand la commune seul porter le projet et que l'intercommunalité ou le département n'intervenait pas, soit que l'étau des marchés financiers à l'époque était trop élevé, soit que les taux ont ne sont pas des taux fixes et ont explosé avec l'augmentation des taux, notamment lors de la dernière crise financière avec des préfets par des banques étrangères notamment, soit que les travaux de rénovation et les loyers ne correspondait pas effectivement aux arrondissements qui avait été évoqué, je pense qu'il y a pas un modèle aujourd'hui de brigade ou de construction de casernes, il y a des modèles et qu'il faut que nous regardions les modèles qu'ont le plus porter atteinte à la vie des militaires, puisque les collectivités ne faisait parfois même plus les travaux du fait qu'il ne pouvait pas payer des investissements alors nous, nous réfléchissons au ministère de l'Intérieur, il y a d'ailleurs une phrase dans le rapport annexé sur ce sujet, a créé une foncière du point de vue de l'État pour l'ensemble des travaux du mystère, l'intérieur, je dis au ministre de presse en le regardant, c'est une, c'est une idée qui n'est pas neuve, mais qui est intéressant, parce que l'État ne l'a jamais mis en place, ne faut-il pas créer dans des ministères qui ont beaucoup de logements, les militaires de caserne commissariat de, de, de, de, de, de, d'hôtels particuliers des préfectures. Et devant la rénovation énergétique qu'on doit mettre en place, et aussi la la rénovation simplement des usages, à commencer par la numérisation, est ce que on n'a pas intérêt à créer une foncière, soit c'est une frontière propre à la police nationale, une à l'ATE admiration préfectorale et une gendarmerie nationale soit une commune au ministère de l'Intérieur, soit une commune pour tout l'État peut tout à fait imaginer que l'État créer sa foncière mais plus on a agrandit évidemment les acteurs, plus c'est complexe et technocrates. Tic, donc faisons ça peut être au niveau d'abord du ministère de l'Intérieur et singulièrement de la gendarmerie nationale qui sans doute ah les difficultés d'immobilier les plus importants parmi toutes les administrations, que j'ai l'honneur de diriger à la fois pour répondre à l'interrogation de ce rapporteur notamment sur les montages financiers qui l'évoquait à la fois pour répondre à votre interrogation, c'est-à-dire les loyers qui correspondent pas forcément à la le nombre de familles qui a, qui habite dans dans ses casernes et à la fois pour répondre aux objectifs d'accueil de modernité de énergie distribuée négativement, si j'ose dire, et donc la création de cette foncière, je pense qu'il faut modifier le décret que vous évoquez, donc j'apporte pas de réponse définitive à vos interrogations, je trouve aux pistes de réflexion intéressante et j'adopte, si j'ose dire, bien volontiers une position d'acceptation de de vos amants de vos amendements je terminerai par dire mesdames et messieurs les sénateurs que la difficulté que nous avons c'est que nous utilisons sans doute pas assez lorsqu'on en responsabilité locale d'autres moyens que la loi permet tout à fait utiliser par exemple les bailleurs sociaux. Il est tout à fait possible de se retourner dans son bailleur départemental et de lui dire : voilà, j'ai une caserne de gendarmerie que le ministère va m'octroyer parce que j'ai voté la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, c'est une façon pour le département où l'intercommunalité qui porte ou parfois le 1 % logement, enfin en tout cas les bailleurs privés, qui peuvent aussi tout à fait intéressé à l'histoire, vous construisez l'école la brigade de gendarmerie, le logement des militaires qui, en général mieux construit que quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait et par ailleurs, vous faites votre propre le développement urbain que vous souhaitez à l'échelle du village où, chef d'une petite ville, on utilise aussi peut être pas assez facilement les dispositions notamment que les bailleurs sociaux peuvent nous offrir, surtout lorsqu'il s'agit d'équipements publics comme les gendarmeries quelques-uns le font, mais c'est vraiment pas la majorité du jour pour prendre l'expression du film, donc vraiment on est très ouvert, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Merci Madame Goulet. vous avez été particulièrement bienveillant sur ce dossier, le dossier de la gendarmerie Tourouvre sur hein, parce que là les, les chiffres sont sensibles : 1 50 1000 euros, le ministère de l'Intérieur 193000 les loyers sont vraiment trop bas, mais je voudrais aussi dire que de nombreux efforts ont été faits, car désormais ce type de construction peut bénéficier du FCTVA ce qui n'était pas possible avant l'année dernière, la loi de finances désormais le permet donc le retour du FCTVA est quand même aussi très important, ça, ça crée évidemment une grosse différence dans le dans l'économie de la construction, mais en toute hypothèse, monsieur le ministre il est, il est certain que les loyers sont en général trop faible, ceux qui sont payés en tous les cas, par le ministère de l'Intérieur, sont en général trop faible pour assurer l'économie quoi qu'il en soit, je crois que le cas de la gendarmerie Tourouvre est réglée grâce au préfet, qui a été tout à fait à l'écoute des habitants qui avait besoin de cette gendarmerie je pense que cet amendement est extrêmement bienvenu et en tous les cas je le voterai. Merci madame Gisèle Jourda merci madame la présidente. Simplement dire bien entendu que je suis extrêmement favorable à ces amendements et notamment celui que nous avons donc présenter avec Philippe Paul pourquoi parce qu'il y a une heure et les interrogations sur nos territoires par rapport aux collectivités locales, alors cela se pose tant de pneus milieu rural que local, le milieu péri-urbain parce qu'on a tellement fermé incertaine au moment tellement redéployer qu'on a plus

et je suis tout à fait, j'ai été sensible aux propos de Monsieur le Ministre, lorsqu'il dit qu'il faut adapter parce qu'effectivement la vie des gendarmes a chargé, et nous nous devons de faire et de proposer quelque chose qui soit cohérent lorsqu'on voit les parcs que nous avons de logements avaient l'obligation des gendarmes d'y être et comment ils ne répondent plus aux objectifs de la vie moderne, telle que nous la concevons et de la dignité même hein, il y a, il y a certaines logement vous parliez monsieur le Ministre des bailleurs sociaux, mais à un moment, il y a la rénovation de ses locaux, donc je crois que là, avec le vote de de de cet amendement, cet homme, un 1er pas et surtout ça crédibilise ce projet des 200 brigades supplémentaires qui répondent un maillage territorial. Merci monsieur Rickman. Merci madame la présidente, oui, Monsieur le Ministre, c'est pas tant la volonté de faire des gendarmeries, c'est surtout qu'il faut que les dossiers aboutissent, vous êtes venus en Haute-Saône, l'année dernière, posé la première Pierre de la gendarmerie de champagne et il y a 3 projets de gendarmerie en Haute-Saône, champagne et j'essaye d'empire sur Salon le dossier qui a été lancé le plus récemment date de quasiment 10 ans on a trouvé les systèmes hein agissait on a mis à disposition un terrain, on a fait un appel d'offre un constructeur privé sous condition qu'ils construisent une gendarmerie c'est Habitat 70 le bailleur social qui a obtenu le marché il y a bientôt j'étais encore maire il y a bientôt 4 ou 5 ans, le permis va peut être être seulement déposé fin d'année, donc je pense que non seulement, faut avoir la volonté de construire des gendarmeries de toute façon, on ne peut pas faire autrement, quand je vois les bâtiments de la gendarmerie de Jussey aujourd'hui, on est à la limite de l'insalubrité, faute de moyens, faute de travaux, mais c'est surtout que ces dossiers sont très, très, très long et et il y a tellement de conditions tellement de de grains. De sable dans l'engrenage qui bloque pour 6 mois pour sept mois à chaque fois la la la la la mise en place à la discussion autour du loyer qui va être demandées par le bailleur social à la gendarmerie, les conditions d'urbanisme et pourtant on est sur des projets d'intérêt général et cetera, et cetera et ses dossiers tout sans une lenteur et à chaque fois on dit aux jeunes gendarmes qui arrivent, vous inquiétez pas, vous pouvez rester dans un an, dans deux ans vous aurez une belle gendarmerie mais seulement ça fait longtemps que les premiers qui sont arrivés sont partis et sont dans d'autres brigades que la construction de la gendarmerie n'a pas encore débuté, je pense que c'est un des points très importants, c'est le fait de se donner la possibilité d'accélérer les dossiers merci. Merci monsieur la Mini. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, Monsieur le président de la commission des lois, messieurs, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, c'est c'est important d'aborder ces ces sujets, les collègues qui sont sont exprimés l'ont rappelé et je crois que le volet humain, il est fondamental, les moyens humains, au niveau, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, etc, mais pour les casernes de, de gendarmerie et Monsieur le Ministre, en en début d'intervention, cet après-midi, vous l'avez rappelé parce que je dirais les les gendarmes et leurs familles habitent et travaillent aussi sur place, c'est différent, des policiers et et historiquement, je dirais les les casernes, moi je prends l'exemple de des Ardennes, que je connais bien les les casernes, c'est principalement des propriétés départemental et encore quelques quelques casernes, c'est l'État qui en est propriétaire et je pense que, à ce niveau-là, bon, c'est compliqué, il faut le reconnaître, il y a toujours des travaux à faire, d'entretien, de maintenance, il y a eu quelques casernes constructions neuves récemment ces dernières, ces dernières années mais la tâche reste immense, parce que je dirais,

2 budget qu'on met de l'argent, et quand on met de l'argent peut rénover bien sûr là on voit les voitures et tout le monde sait par nous qu'on a des commissariats des casernes vétustes, on n'a pas fait par en un jour, il ne fera pas la réduction d'un jour, par contre, avec une progression que nous autres ensemble pourront faire demain matin on va rattraper le retard et je crois que on parle tous unité votons les Budgets nécessaires au ministre pour pouvoir effectuer ces travaux. Merci, alors je vais mettre aux voix, donc ces trois amendements identiques 23 211 225 avis favorable de la commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient sont donc adopté amendement 215 Monsieur Mohamed soit élu. Oui, madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, les faits divers tragiques se multiplient et un deuil, les familles en outre-mer augmentation record des homicides par arme à feu et arme blanche recrudescence des braquages, violence liée au trafic de drogue féminicides violences contre les forces de l'ordre, l'insécurité grandissante gagne toutes les catégories sociales des annonces ont été faites pour endiguer cette insécurité en outre-mer, avec le déploiement de nouveaux moyens humains et matériels en 1er lieu déployés aux frontières des Outre-mer de nouveaux outils technologiques pour lutter contre les trafics avec des scanners aurait eu pour bagages des scanners corporels des scanners à conteneurs dans les grands ports des moyens nautiques des radars de surveillance ensuite en matière de lutte contre la délinquance et de protection de leur public, les outre-mer bénéficieront de l'augmentation des effectifs de gendarmes départementaux de réservistes et d'unités de forces mobiles supplémentaires aussi l'implantation de nouvelles brigades de gendarmerie nationale telle que proposée par La Lopmi est une mesure rassurante pour restaurer l'ordre républicain dans ces territoires, à ce titre, et au regard de la dégradation inédite du climat sécuritaire et de nos spécificités, le présent amendement prévoit une attention particulière dans le choix d'implantation de nouvelles brigades en outre-mer. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, j'avais demandé de la même manière que un autre amendement précédent qu'on rectifie à la rédaction pour qu'elles s'intègrent mieux dans le texte d'orientation, c'est légitime qu'on pose ce problème de spécificité des outre-mer, en plus, on a un ministre qui est de l'Intérieur et des Outre-mer et qui connaît bien, c'est cette question donc rectifier tels favorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. comme ministre des Outre-Mer et de l'Intérieur, monsieur le rapporteur, donc je peux donner qu'un avis favorable, oh la la, la maman du du sénateur Tani Quelques mots quand même sur la spécificité ultramarine qui repose aussi sur une population devenue très importante dans les zones gendarmerie c'est aussi une difficulté que nous avons à à Mayotte, mais nous avons dans doute ta étant la République mais quand même singulièrement à à Mayotte et que si il y a bien un endroit où la question en zone police et gendarmerie se pose, c'est bien dans les territoires ultramarins régulièrement ceux qui connaissent une augmentation de population en même temps qu'une augmentation de délinquance, donc je voudrais vraiment dire que c'est pas simplement une pétition de principe au fait pour vous plaire, monsieur le sénateur, et qu'effectivement nous devons regarder des implantations supplémentaires en mer, vu la délinquance plus fort, ce qui s'y trouvent, j'ai fait des annonces sur la Guyane où j'ai annoncé 4 brigades de gendarmerie parmi d'autres annonces je reviendrai vous le savez, à Amélia, toujours à l'occasion effectivement de pouvoir annoncer 4 nouvelles brigades également dans votre département, je n'avais pas fait jusqu'à présent, mais je vais vous le dire parce que vous avez fait cette sollicitation et que ces quatre, brigade de création à à Mayotte, si nous pouvons trouver des des très rapidement à un endroit pour y implanter les militaires de la gendarmerie sont disponible dès l'été prochain. Merci, alors je vais mettre aux voix l'amendement 215 qui a reçu un avis favorable de la commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il est donc adopté l'amendement 156 messieurs faire nickel. Oui, madame la présidente, monsieur le Ministre, chers collègues, cet amendement propose de de renforcer et généraliser la possibilité de cette mutualisation intercommunal des gardes champêtre, qu'on appelle en Alsace brigades vertes, en effet, depuis 1988 en s'appuyant particulièrement sur la spécificité, la spécificité de notre droit local, donc la forte densité des gardes champêtre en Alsace Moselle, un amendement du sénateur Goetschi, a permis cette dynamique qui a commencé dans le Haut-Rhin, avec une cinquantaine de communes aujourd'hui c'est plus de 370 et ça a débordé sur le Bas-Rhin donc la brigade verte constitue une garantie de protection des milieux naturels de la faune, de la flore flore sauvages sur les territoires des communes qu'elle couvre, contribuant à réduire drastiquement les incivilités dans les milieux naturels et la porte par ailleurs un appui aux agriculteurs en contribuant à réduire les vols l'organisation répond aux besoins des communes et les coûts sont répartis le conseil départemental donc maintenant la collectivité européenne d'Alsace en prenant une part importante. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Alors j'invite Monsieur faire à à relire quand même les les débats du Sénat parce que nous en avons parlé longuement dans la loi sécurité globale à l'initiative du Sénat, nous avons donné la possibilité de mutualiser un garde champêtre entre plusieurs EPCI, c'était dans la loi ah engagement et proximité en 2000 19 et le Sénat s'est à plusieurs reprises prononcé pour la fusion du Cadre d'emplois des policiers municipaux, des gardes champêtre, donc sur l'intention tous les travaux du Sénat vont dans le sens de cette mutualisation et et de fusion de 2 Cadre d'emplois sauf que telle qu'que rédigé l'amendement de généralisation, c'est une atteinte évidente à la libre administration des collectivités locales, et je ne peux qu'être défavorable. donc je mets aux voix l'amendement 157 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 158 Monsieur faire Cet amendement donc vise à permettre aux gardes champêtre d'avoir recours aux moyens technologiques modernes tels que les appareils photographiques dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux propriétés rurale et forestière dépôts sauvages en milieu naturel vole dans les champs, sur les exploitations agricoles et ce afin d'établir la réalité de l'infraction.

Merci madame la présidente, cet amendement qui est demandée par plusieurs plusieurs intercommunalités vise à élargir le périmètre des agents pouvaient être pouvant être assermenté en matière de police des déchets à de nombreuses reprises en 2014 comme en 2020 les maires et présidents d'intercommunalités ont fait obstacle au transfert de de police administrative, non pas au motif que cet objectif n'était pas souhaitée et parce que le juridique actuel complique l'effectivité des décisions prises par les présidents auxquels sont transférer ses pouvoirs de police, ceci est particulièrement marquée pour les attributions correspondant, domaine de la collecte des déchets et la gestion des déchets sauvages, en effet, le code de l'environnement restera la liste des agents qui peuvent être assermenté pour procéder à la recherche et la constatation des infractions à la matière sont visés, notamment des agents qui ne sont pas employées par les collectivités locales, agent des douanes, de la répression des fraudes ou ne le ne le sont ne le sont que par celles qui dispose d'importants moyens, agent de police judiciaire adjoint médecins territoriaux sans modifier donc le code de l'envie de roman le présent amendement permet au présent, présidents d'intercommunalités en complément des possibilités d'ores et déjà prévues par ce code de missionner d'autres agents spécialement assermentés pour rechercher et constater les infractions au règlement établi et, le cas échéant en matière de collecte des déchets et de déchets sauvages merci. Merci la vie de la commission, monsieur le rapporteur. Là encore, ce débat a eu lieu à plusieurs reprises ici au Sénat, et notamment au cours des lois de décentralisation ma ma ma très estimables collègues Françoise Gatel qui préside notre délégation collectivités locales à une formule laissons l'Intelligence territoriale jouer son rôle et les acteurs locaux exercer leurs compétences plutôt que d'imposer autoritairement de transférer des compétences des communes vers l'intercommunalité, parce que ce n'est pas justifiée dans tous les territoires défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Je ne saurais dire mieux que le rapporteur de presse se cependant, je voudrais quand même remarquer que cette possibilité a été adopté lors de la loi climat et résilience ce 22 août 2021, c'est l'article 293 de cette loi que vous avez, je crois, voté dans cet hémicycle. Merci monsieur le président Gontard. Ben du, du coup, je vous invite à relire l'amendement parce que il ne s'agit pas du tout de ce que dit monsieur le rapporteur, ni ce qui a été effectivement adopté dans dans la loi, dans la loi climat on a de nombreux présidents d'intercommunalités en fait c'est juste donner la possibilité, il y a aucune obligation et, bien sûr que c'est la liberté de chaque collectivité mais juste de pouvoir assermentés ces ces, ces, ces délits, donc c'est assez simple, hein, et c'est ce qui bloque un certain nombre de collectivités et de l'intercommunalité et je suis prêt à en parler avec Madame, avec la sénatrice Gatel d'ailleurs pour qu'on puisse avancer sur cette sur Merci, alors je mets aux voix donc l'amendement 158 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 200. madame Gréaume. Merci madame la présidente, notre amendement vise à supprimer dans le rapport annexé le postulat erroné selon lequel la procédure pénale serait une lourdeur inutile, alors que l'état un ensemble de droits par pour les citoyens, il convient en outre de souligner que la modification de la procédure pénale, Champ de compétence propre du ministère de la justice n'a pas sa place dans une loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, merci. Je suis d'accord avec Madame Assassi sur les 2 points mais ça n'empêche pas de mentionner ces points dans le rapport annexé tout l'enjeu, la, la, la réforme de la procédure pénale et de l'alléger pour que les policiers, gendarmes, sans affaiblir la protection des droits, libertés soit plus sur le terrain, je vois pas ce que on devrait supprimer dans un rapport qui indique une orientation claire défavorable. Merci l'avis du gouvernement, mais ma vie merci je mets donc aux voix l'amendement 206 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour, qui contre qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 101 monsieur Bena Roche. Madame la présidente, merci, alors que le gouvernement en fait présente dans cette loi pacte citoyen de confiance nécessaire et légitime de la population envers l'ensemble de ses forces de sécurité, je pense qu'il convient de garantir clairement la possible l'identification des acteurs de la sécurité dans l'exercice de leurs fonctions, notre commission a décidé de de pas soutenir cet amendement en ce qu'il serait satisfait. Mais une fois encore, cet amendement cherche à inscrire dans le cadre d'une loi de programmation donc des prochaines années, les axes essentiels qui sont, qui sont ceux du ministère de l'Intérieur et parmi ceux-ci, nous pensons que celui de l'identification anonymisé des forces de l'ordre en état et doit y figurer si la visibilité de la carte professionnelle des agents de la police municipale étude obligations garanties par le code de sécurité intérieure, celle-ci doit être complété par le but recherché, à savoir l'identification de tous ceux qui garantissent la sécurité des citoyens, cette mesure est un premier pas fort dans la reconstruction de IA solide de confiance entre les forces de l'ordre et les citoyens, nous souhaitons que ça t'identification des agents fasse partie de la culture du ministère de la, de l'intérieur cette identification est un facteur de confiance des citoyens envers leurs poulies. Ainsi l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Pour une fois, monsieur Bena Roche et pour les contrôles d'identité, sauf que ça existe déjà dans l'article R 434 15 du code de la sécurité intérieure et qui satisfait de sa préoccupation défavorable. Monsieur le Ministre, défavorable, donc je mets aux voix l'amendement donc son hein, qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il n'est donc pas adopté 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 178 madame Gréaume. Alors notre amendement vise à supprimer dans le rapport annexé la sous-section de trois intitulé l'objectif de doublement de la présence des forces de l'ordre sur la voie publique, un poste d'activer un ensemble de leviers complémentaires : les dispositions prévues à ces alinéas consacrent notamment la préférence de la compensation financière des heures supplémentaires au jour de récupération en vue de l'ouverture d'une discussion sociale sur l'augmentation du temps de travail au sein des forces de sécurité intérieure, demandé par le président de la République, la mise en place de la fonction d'assistant de police et de gendarmerie et lors l'abandon de tâches périphériques, nous considérons que la préférence de la compensation financière des heures supplémentaires au jour de récupération et l'ouverture d'une discussion sociale sur l'augmentation du temps de travail au sein des forces de sécurité intérieure est une fuite en avant libérale qui casse les droits sociaux des policiers et Brad les services publics La Lopmi envisage de doubler la présence des forces de l'ordre sur le terrain d'ici 2030, via notamment la suppression de missions périphériques mais alors qui s'occupera notamment du transfert de détenus, l'administration pénitentiaire, déjà surchargés de même mettre en place la fonction d'assistant de police et de gendarmerie n'est pas un gage d'efficacité, la procédure pénale, même son aspect le plus infime nécessite vigilance et rigueur merci. marqueurs de l'action sécuritaire qui a été menée sous la la présidence du président justement de la République, Nicolas Sarkozy, la politique du chiffre a été fortement critiquée par les représentants des personnels, gardien de la paix principalement en terme d'efficacité pour lutter contres les sécurités mais aussi en raison de la pression qui a été mise sur ces policiers de terrain qui était conduit à se focaliser sur les statistiques plutôt que sur la délinquance pour les représentants des policiers, il s'agit davantage d'une politique d'affichage et de communication qu'une lutte réelle contre la délinquance, conduite au détriment de la santé, des policiers l'usage renforcé des indicateurs chiffrés pour mesurer et piloter l'activité policière que le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer veut continuer à mettre en avant, c'est pourtant révélé comme l'un des raisons des dysfonctionnements des services de police, en outre, Monsieur le Ministre, comme vous le savez, de nombreux de nombreux social de sociologue, spécialiste des questions de police montre les limites de ses simple bilan chiffré et nous invite à varier l'utilisation de ces chiffres, par exemple en utilisant des expérimentations, ou des modélisations comme cela est fait au Canada ou au Royaume-Uni, il convient donc de rappeler dans le rapport annexé que la mesure statistique de l'effectivité de l'action policière qui va accompagner le doublement de la présence des forces de sécurité sur la voie publique, dans les 10 ans ne peut se limiter à la seule communication du relevé chiffré de l'activité policière dans les médias, sachant que ceux-ci ont aussi subissent des effets de conjoncture ou des variations dans le temps des thématiques. Si Monsieur Bénard Roche pour le d'en finir mais d'avancer à rythme non forcé dans le tout numérique et le tout distanciel que par ailleurs je rappelle notre assemblée n'aime pas terriblement puisque même en interne, nous avons décidé de terminer avec les visio pour les réunions de commissions peut avoir un avis différent là-dessus mais enfin en tout cas, c'est ce qui a été décidé. Le rapport annexé lui annonce que des actes d'enquête et les audiences du juge des libertés et de la détention, notamment pour les auditions de placement, c'est en en craint en centre de rétention administrative semaine rend en priorité. Par voie de communication audiovisuelle quand on a visité Dekra et quand on est allé voir les JLD qui étaient à côté par exemple à Marseille je pense pas que ce soit une mesure qui amène un n'enthousiasme démesuré d'aucune des parties de ces audiences parce que les audiences en fait qui sont, qui aurait été très développé depuis la pandémie du Covid ne permettent pas en fait d'assurer pleinement ni la confidentialité des échanges entre les parties et et leurs avocats, ni la solennité des audiences qui est fortement réduite lors des procédures par écran interposé, elle est décriée comme je vous l'ai dit, et je l'ai constaté dans plusieurs gras et c'est plusieurs JLD par plusieurs professionnels de la justice tant avocat que magistrats et elle illustre en fait un sorte de sorte de choix du gouvernement de développer une justice alors si, si on est gentil, on va dire, plus, plus rapide et si on est moins gentil, on va dire un peu expéditive au détriment du droit des justiciables généraliser cette pratique conduit en fait à porter atteinte à la qualité de la justice rendue et nous assistons déjà une dégradation progressive des audiences en matière de droits des étrangers en France concernant les actes d'enquête si ces dernières heures, les enquêtes applique la participation de justiciables, il convient pour nous de matières systématiquement une présence physique des agents pour les usagers qui ne souhaite pas réalisé les actes par voie de télécommunications audiovisuel. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur, sur ces trois amendements. Alors, le ministre a dit à juste titre, c'était une forte attente que il voulait doubler la présence des forces de l'Ordre sur la voie publique, le moins qu'on puisse attendre d'un rapport d'orientation, c'est qu'il explique les modalités qui vont permettre de doubler les forces de l'Ordre sur la voie publique, il y a donc une série de précision dans le rapport d'orientation qui sont tout à fait pertinente, et donc je ne peux quatre défavorable au numéro 178 de Madame Assassi, de même que celui de Monsieur Durand, parce qu'il faut bien avoir des chiffres pour le vérifier, et celui, 74 de Monsieur Bénard, Roche, parce que l'objet de son amendement, c'est de maintenir systématiquement une présence physique des agents pour les usagers qui ne souhaite pas réalisé les actes par voie de télécommunications, alors que quand on fait des audiences télé à part par les voix de télécommunications toutes les garanties sont apportées pour en particulier pour les étrangers, avec les moyens de télécommunications audiovisuel la confidentialité de la transmission, tout cela est donc déjà réalisés et c'est normal que le rapport explique les modalités qui permettent d'atteindre un objectif défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. merci à la présidente : j'avoue pas vraiment comprendre les amendements de suppression. En tout cas si de suppression du fait que oui je je parle madame Assassi en tout cas de son groupe. Parce que. Je ne vois pas en quoi. Mettre plus de policiers, de gendarmes dans la rue et donc accepter ce que une grande partie de la gauche ne propose, c'est-à-dire une police plus présente. Moins d'interventions et plus d'accompagnement de de présence qu'on pourrait qualifier de proximité en soi, la police en soi, elle doit être de proximité est une fuite en avant libérale j'ai du mal à suivre puisque ce que nous évoquons ici dans cette démonstration, c'est que par une augmentation d'effectifs que vous êtes très nombreux à me demander quels que soient les groupes politiques par la réserve opérationnelle. Par un certain nombre de suppressions de tâches périphériques, j'y reviendrai, on utilise policiers et de gendarmes pour faire ce qui ce pourquoi ils sont engagés, c'est-à-dire pour être présent sur la voie publique, alors Madame la cerise dites qui va s'occuper des instructions judiciaires bah oui, l'administration pénitentiaire, de même qu'il est normal que les policiers s'occupent de la délinquance alors est-ce qu'ils ont assez de moyens pour le faire, ça c'est une question intéresse. Hier, non demain oui dans le PLF que vous allez voter il y a 200 équivalents temps plein, qui ont été prévu puisque nous avons fait un rapport avec le ministère de la justice, créée il y a 200 agents de l'administration pénitentiaire, créé pour justement remplacer les policiers qui, dans toutes les villes de province notamment, prennent deux 3 personnes dont une patrouille pour aller faire de l'extension de la maison d'arrêt pour présenter devant le juge. Ou l'extraction du commissariat pour le présenter à la maison d'arrêt et c'est pas le travail des policiers que de faire ce travail, en soi c'est ça n'a aucune avancée policière que le faire ce qui est vrai c'est que nous avons, nous, au ministère de l'Intérieur depuis de très nombreuses années suppléer au manque de moyens du ministère de la justice, mais en attendant, ça veut dire que dans une ville qui connaît un tribunal correctionnel, quand il y a 4 patrouilles dans la journée, ben ça veut dire qu'on a deux qui sont occupés à faire extras judiciaire et pendant ce temps,-là, ils ne sont pas en train de répondre au dix-sept ou en train de faire des patrouilles dans le centre-ville ou dans les quartiers populaires, donc il c'est pas une fuite en avant libérale niveau, vous ne voyez pas d'ultra libéralisme partout, il y en a déjà assez, me semble-t-il, de dire qu'il faut qu'il y ait plus de présence voit policiers là franchement je ne comprends pas, il y a des moments, je peux comprendre le raisonnement politique du du groupe communiste, je pense, je pense, je pense que vous commettez une erreur d'analyse. Si les assistants d'enquête là aussi je ne comprends pas très bien votre sujet d'ailleurs, je vais vous dire vous vous n'avez pas discuté que syndicats qui s'occupe de ces sujets du personnel ministre hâtif parce qu'ils sont tous extrêmement favorable, quelles que soient les syndicats et les quelques-uns qui je pense ne sont pas très éloigné pour bien les connaître de votre orientation politique madame la présidente, je ne vais pas les citer ici mais ils se reconnaîtront, et moi je, je, je, j'apprécie particulièrement, façon de se battre pour ses ouvriers, administratifs qui ne sont pas toujours reconnus par les ministères et notamment par le ministère de l'Intérieur et je veux leur dire ici que le personnel administratif, technique et scientifique, ils font partie de la communauté de la police nationale la, les 3 syndicats qui s'en occupe, sont tous les trois extrêmement favorable à cette réforme et que c'est justement parfois une partie de la police statutaire ou la gendarmerie statutaire qui n'est pas très favorable à cela, je pense que au contraire ça va très largement dans ce que vous essayez de porter dans la fonction publique, c'est-à-dire la montée en en formation en gamme en promotion de personnes qui sont considérées comme des catégories, ceux des catégories B qui, pourtant, connaissait la difficulté que les policiers parfois connaissent des attentats terroristes, on l'a vu avec Madame enfermé à à à Rambouillet et qui vont avoir une compétence particulière, il s'agit pas d'ultralibéralisme, je vous ai pas dit qu'on allait embaucher des contractuels et condamné embaucher des sociétés privées pour le faire, ce sont des fonctionnaires qui ont le statut de fonctionnaire du personnel Misratis du ministère de l'Intérieur,

je pense que là aussi c'est une petite me semble-t-il, incompréhension collective. La politique du chiffre consiste en quoi. Consiste à fixer à des services des objectifs chiffrés de réussite. Par exemple, nous devons baisser de 5 % la délinquance en Saône-et-Loire où je demande à direction départementale de ses de faire 150 AFD dans le mois, ça, c'est la politique du chiffre. Ce n'est jamais ce que j'ai demandé aux services de police et encore moi ce que je demande maintenant ce que je demande aux services de police et ce que je rends public mais comme tous les ministre de l'Intérieur, bon, comme tous les ministres du groupe public rende publiques les chiffres du déficit ou de dépenses publiques et comme tout le ministre du Travail, rend les chiffres du chômage, ses parents, soit un objectif c'est une statistique, elle vaut ce qu'elle vous, vous avez raison, il y a des billets statistiques comme partout mais c'est vrai dans tous, y compris sociologues ont dévié statistiques aussi comme tout est subjectif, par définition, il peut y avoir aussi un certain nombre de de discussion d'un certain nombre de théories et bien sûr, je suis tout à fait ouverts aux analyses scientifiques et et de l'ensemble de ceux qui réfléchissent à la police nationale, la gendarmerie nationale. Mais quand je rends public des chiffres de la délinquance comme tous mes prédécesseurs que ben comme tous mes futurs successeurs je ne fais rien d'autre que révéler l'activité des services notamment les plaintes déposées dans les commissariats ou les interpellations en fait de trafiquants je n'aimais pas d'objectif, je le constate, ce serait d'ailleurs absurde que j'avais des objectifs dans des choses aussi non mesurable au sens police du terme que les violences. J'ai J'ai tendance à penser que dans les chiffres des violences intrafamiliales augmente, c'est à la fois un drame pour ceux qui les subissent, mais en même temps le révélateur que les services de police et de gendarmerie de transforme plus en main courante, ce qui était hier en plainte donc ce n'est pas ça non plus, la politique du chiffre mais par parallèlement Monsieur sept heures, pardon de vous dire que c'est pas anormal que intérieur explique comment, comme l'a dit monsieur le rapporteur, on va réussir à doubler la présence de policiers, de gendarmes sur la voie publique, sinon ce serait un voeu pieux. Et je vous expliquerai ben voilà, on va doubler la présence va publier, je me rassurer et puis vous me direz : ben alors cher ami, comment vous faites. Je l'ai expliqué ailleurs je veux bien leur expliquer 8500 effectifs supplémentaires, cela contribuera à plus de présence de la voie publique. Réserve opérationnelle créés dans la police nationale et nous avons désormais décidé de geler les crédits de réserve qui était auparavant annulé annulé de la gendarmerie nationale, la réserve contribue la présence de voie publique fin des cycles horaires qui prenait trop d'énergie, si j'ose dire. Pour ne pas être sur la voie publique, c'est ce qu'on disait que le sénateur Dominati notamment la fin du vendredi, fort de la police. allégement des procédures pénales, les assistants d'enquête ou les AFD évidemment, vous avez le droit de les combattre, mais ça fait partie de la simplification qui créé plus de présence sur la voie publique quand j'évoqué la démonstration avec le téléphone tout à l'heure, ça fait gagner de la voie publique, enfin des extractions judiciaires

au doublement de la présence de voie publique, n'y voyez pas de shit de chiffres statistiques, j'essaie de justifier devant le Parlement des crédits budgétaires, c'est-à-dire la peau des Français que j'espère que vous allez m'accorder de toute façon, je suis obligée de justifier devant la Cour des comptes, donc il faut quand même qu'on ait des mesures de chiffres, sinon on aurait un débat 20, 20, voyez ce que je voulais dire, Monsieur le Sénateur, donc il n'a jamais été question depuis que je suis ministre de l'Intérieur et je crois que c'était vrai de mes prédécesseurs également de donner à des chefs de police des réussites en pourcentage d'affaires, ça ça amène effectivement à pas prendre des plaintes à transformer en main courante, on va dire à des gens, on prend pas votre plainte dans un commissariat pour essayer de faire baisser les chiffres où ça fait perdre du temps aux procédures pour que d'une année sur l'autre côté de procédure novembre on ne arrête pas avant janvier pour montrer que le ministre de l'Intérieur avait raison donc je suis tout à fait d'accord ça c'est pas possible, en revanche, qu'on dévoile les chiffres de la délinquance, ça me paraît normal qu'on en discute, y compris pour vous expliquer pourquoi ça augmente, pourquoi ça baisse et qu'on ne soit pas d'accord sur le constat et quand on n'explique comment on arrive à doubler, ce qui est un effort considérable, la présence de voie publique cent doubler le nombre d'effectifs de voie publique. Ben je pense que ça demander une démonstration, donc je suis vraiment pour qu'il y ait pas de, de, de difficultés de compréhension entre nous, il s'agit, pas dans les dispositions que je vous présente, pour ceux qui n'ont pas le texte sous la le, le, la main de revenir à une politique du chiffre qu'évidemment je ne comprends pas non plus dans mes actions politiques.

Merci madame la présidente, cet amendement vise à supprimer dans le rapport annexé la présentation de la simplification de la procédure pénale comme levier pour renforcer la présence des forces de l'ordre sur la voie publique, outre l'identification erronée de la procédure pénale à une lourdeur inutile alors qu'elle est un ensemble de droits pour les citoyens. Nous considérons donc faire de la simplification de la procédure pénale, une priorité, c'est prendre le risque de faire fi des gares Andy procès du Real qui procédurale qui entoure la garde à vue notamment, et cela ne va pas dans le sens de la valorisation des métiers de la sécurité intérieure, abaissant les exigences qui entourent ceci et qui donne du sens au travail de la police judiciaire. la lourdeur de la procédure pénale, allez, d'une part parce qu'il y a un certain nombre de garanties et de droits qui sont préservés grâce à cette et peut être rigidité parfois excessive, mais aller aussi parce qu'il y a des tas de de de systèmes, dans le cas de cette procédure, qui sont sur superfétatoire alors certes ça relève d'une d'une réforme systémique de de la justice qu'on attend comme soeur Anne depuis longtemps après les états généraux, mais d'un autre côté, on on ne peut pas empêcher un autre ministre, pour ce qui le concerne de détailler par exemple, il nous a expliqué les réquisitions certains nombre de choses de ce type, et donc il y a un certain nombre de choses qui en allégeant cette procédure permette de remettre dans d'enlever des tâches administratives superfétatoire et de remettre des policiers sur le terrain, donc avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement, même avis merci donc je mets aux voix l'amendement 205 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté cet amendement faisant l'objet d'une discussion commune le cent 80, monsieur Laënnec. Merci madame la présidente, cet amendement vise à supprimer dans le rapport annexé la sous-section de quatre intitulé je cite maître la victime au centre de l'attention cette sous-section du du rapport envisage de refondre le parcours de victimes depuis l'accueil jusqu'au suivi de plaintes en privilégiant la dématérialisation de plus cette sous-section met l'accent sur une prise de plainte hors les murs, accompagnons accompagné d'un traitement rapide et l'expérimentation de l'utilisation d'un robot d'accueil, nous rejetons la dématérialisation du dépôt de plaintes et de son suivi une prise en charge des plaintes hors les murs et hors de propos et instaure de fait une distance qui ne devrait pas avoir lieu entre victimes et police

qui sont formés sur des thématiques, elles étaient LGBT phobies alors elle demande parce que ça existe déjà dans un certain nombre de villes par exemple à Bordeaux et à Paris. ils sont chargés dans ces villes de recevoir les plaintes et de traiter les procédures liées à l'homophobie à la transphobie, ils sont également en charge de former leurs collègues sur les violences homophobes ainsi il pourrait permettre d'unifier les prises en charge des victimes d'homophobie sur l'ensemble du territoire c'est Jason de liaison permis dans les territoires dans lesquels ils sont déjà implantés, une augmentation du taux de plaintes des victimes d'acte homophobe ou transphobe alors j'ai j'ai entendu le le le les rapporteurs me dire lors de l'examen en commission, après tout, pourquoi que LGBT plus et pas pour d'autres populations fragiles, je vous dis, chers collègues, chiche, notre groupe vous prend au mot nous voterons favorablement tout amendement ou sous-amendement qui visera généraliser la mise en place d'officiers de liaison pour des victimes ou de population fragile voilà, d'autant plus que 2 officiers ont prouvé leur intérêt et leur efficacité dans la prise en charge des victimes et dans leur accompagnement là où ils sont en place. Merci madame la présidente, c'est un amendement de ma collègue Mélanie Vogel, qui vise à un meilleur accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles, alors que, une jeune femme sur 5 serait concerné par le cyber sexisme à caractère sexuel, nous vous proposons donc de l'enregistrement audiovisuel du dépôt de la plainte et d'épreuves en rendant accessibles ces enregistrements aux victimes, vous vous imagineriez répété 7 ou 8 fois lors d'une procédure devant des personnes non formées à ce que vous avez traversé qu'on a volé des photos nues de vous et qui circulent en ligne et que vous vous êtes publiquement harcelés,

d'autres mesures permettraient un meilleur accueil des victimes avec notamment la présence de spécialistes formés sur ce sujet et la présence d'une avocate ou d'un avocat lors du dépôt de la plainte. Il me semble que ses propositions vont dans le bon sens de l'objectif de ce rapport et de son intitulé explicite, il vise à replacer la victime au centre de l'attention et prendre mieux en compte les spécificités. Merci l'amendement numéro neuf Madame rien. Merci madame la présidente, en fait, vous prévoyez dans le rapport des maisons de confiance et de protection de la famille en fait c'est un un nouveau nom d'une d'une chose qui existe et qui est très utile pour prendre en charge spécifiquement les les victimes vous dites une par département et en fait je fais un peu référence aux Maisons France service dont on disait une par canton et dont on se rend compte que ça n'est pas suffisant et donc tout a changé quand on a dit au moins une par canton et là, je voudrais qu'on puisse mettre au moins une par département, de telle sorte qu'on puisse envisager d'en avoir éventuellement au moins une par circonscription. Merci l'amendement 173 madame Carrère. Merci madame la présidente, lors de l'examen du texte par notre commission des lois, un certain nombre d'amendements ont été adoptés afin d'inscrire dans le rapport annexé au projet de loi les objectifs en matière d'accessibilité et d'accueil des personnes en situation de handicap en effet nous ne pouvant que constater le retard que la France accuse en matière d'accessibilité universelle de nombreuses études, le rappelle qu'il s'agisse de l'accessibilité des transports de la voirie, des administrations, des lieux, des espaces dédiés à la santé ou encore au logement des textes sur l'obligation d'accessibilité existe pour autant leur mise en oeuvre reste très limitée et pénalise quotidiennement les personnes hein, situation de handicap, or l'accès au service public est essentiel à l'effectivité des droits des personnes en situation de handicap aussi puisque dans ce projet, le ministère de l'Intérieur souhaite moderniser les locaux des brigades et commissariats pour améliorer la confidentialité et l'ergonomie des points d'accueil le présent amendement vient ajouter un nouvel objectif : la mise en accessibilité de ces, de ces lieux, je vous remercie. Merci l'amendement 73 monsieur Bena Roche. En fait, nous voulons parler maintenant de l'expérimentation de robots d'accueil dans les locaux de police et de gendarmerie Robocop dont on parlait tout à l'heure, entre autres, le livre blanc de la sécurité intérieure publié le 16 novembre 2020, avait fait le constat suivant que nous partageons tous, améliorer la qualité de l'accueil du public et là des vecteurs 1er d'une relation de confiance entre la population et les forces de sécurité intérieure, ces robots d'accueil existe déjà dans certains pays d'Asie et du Moyen-Orient, nous pouvons donc avoir une idée de la façon dont ça pourrait se passer, et en aucun cas, là où ils existent, ils ne représentent une solution pour améliorer l'accueil des victimes, le respect de la confidentialité pour les victimes commencent dès le pré-accueil et l'accueil au comptoir, je, je vous rappelle qu'à ce stade, les victimes doivent financer le motif complet de leur plaide l'attitude d'ailleurs et le nombre de policiers et de policière au comptoir d'accueil favorise ou défavorise déjà reçoit la confidentialité, c'est pour cela qu'un rapport de la préfecture de police de Paris qui a été publié le 3 mars 2019 préconise aux femmes victimes de violences, d'être entendu dans un cadre confidentiel, me paraît un peu incroyable, je dois l'avouer d'expliquer qu'un robot qui ne peut se substituer à un être humain ne saurait exercer des missions d'accueil qui sont très importantes pour le bon déroulement du recueil des plaintes l'accueil représente la première étape de l'accompagnement des victimes qui, souvent, ont du mal à exprimer leur expérience cette expérimentation nous semble au contraire pour voir dégrader très fortement les conditions d'accueil des citoyens qui souhaitent privilégier les relations humaines dans des périodes parfois très difficile de leur vie. Merci, alors l'avis de la commission, monsieur le rapporteur sur l'ensemble de ces amendements. Alors je suis allée prendre parce qu'ils sont de nature diverses, madame la présidente, sur l'amendement 182 Madame Assassi qui concerne essentiellement le développement de l'application ma sécurité que j'avoue que je ne connaissais pas que j'ai chargé sur mon téléphone portable et que je trouve tout à fait télé intéressante et efficace, moi je pense que ça porte amélioration pour les victimes et je suis donc défavorable à ce qu'on supprime ces alinéas sur l'amendement 76 de Monsieur Bénard Roche je pense que le ministre, enfin, il vous dira son ami et tout à fait favorable au développement de la présence d'officiers de liaison LGBT plus d'ailleurs que c'est aujourd'hui dans le déploiement qui se poursuit, progressivement, plutôt une réussite, donc il y a pas de souci là-dessus, mais si vous commencez à le mettent dans un rapport, il faudra mettre d'autres choses dans le rapport enfin et et on l'a, on cible une catégorie de population ça marche effectivement moi j'y suis pas pour principe opposé mais et voilà le rapport telle qu'il est écrit : il faudra mettre d'autre chose derrière, en tout cas c'est sûr que c'est aujourd'hui une première expérience qui est une réussite sur le 131 madame Vogel l'enregistrement des dépositions effectuées par les femmes dans des conditions respectueuses leur intimité, c'est vrai que ça existe déjà pour les mineurs, mais ça paraît moins justifié pour les femmes adultes lorsque plusieurs auditions succède sans principes pour obtenir des précisions et des compléments dans l'enquête, il ne faut pas sous-estimer, par ailleurs, les moyens techniques et les locaux qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre ce principe donc défavorable sur l'amendement de Madame Veil rien moi sur le fond, je pense que c'est plutôt un bon amendement mais faudrait que Monsieur le Ministre, nous donne son avis, puisqu'elle propose qu'à compter de 2024 soit maintenu une maison de confiance et de protection de la famille, dans chaque département, donc je sollicite l'avis du gouvernement, s'il y était favorable, nous y serions également favorable. Sur l'amendement de Madame Carrère qui demande à ce que on renforce les questions d'accessibilité des brigades et commissariats et qu'on aille plus loin et mette ergonomie et accessibilité, ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on a accepté, dans d'autres amendements donc favorable sur l'amendement 73 monsieur Bénard Roche : suppression de la notion d'expérimentation de robots d'accueil dans les commissariats et brigades c'est une expérimentation, évidemment que il ne va pas y avoir des robots d'accueil dans tous les commissariats et qu'on va pas remplacer tous les accueille des commissariats par des robots, enfin, pour être un petit peu, bon c'est il y a certains points d'accueil. Comme, comme dans d'autres services publics d'ailleurs, il y a certains points ou comme dans moi j'ai été maire 29 ans dans certains des établit. Bon, pour les personnes âgées, ça peut être une aide significative mais jamais ça ne va on va remplacer la présence humaine, en tout cas c'est pas ce qui était écrit dans le rapport : avis défavorable.

l'c'est un amendement qui vise à améliorer la, la, la formation des polices spécialisées lors de l'adoption de la loi visant à lutter contre le harcèlement scolaire cette année, le volet pourtant pourtant essentiel de la lutte contre le cyber-harcèlement le cyber sexisme à caractère sexuel, a été exclue du texte, un vraiment que, alors que, une jeune femme sur 5 serait concerné par ces situations, les données nous manque pour l'ampleur exacte du phénomène, mais les conséquences sont dramatiques est réel des jeunes filles mineures se suicide suite à du harcèlement scolaire et cyberharcèlement liée à la fuite de photos de nu qui circule sur des réseaux sociaux et Internet hors collèges et lycées, le cyber sexisme est omniprésent sur nos réseaux et Internet et a un impact sur le bien-être de la sécurité des jeunes filles et femmes. Ces situations nous rappelle que nous devons faire appliquer, comme l'a annoncé le ministre de l'éducation, l'obligation des cours d'éducation à la sexualité au consentement afin d'apprendre l'égalité de genre et lutter contre les stéréotypes et violences sexuelles dès l'école, dans ce rapport annexé vous proposez que la police spécialisée à la protection des enfants puissent sensibiliser les élèves aux violences sexistes et sexuelles et harcèlement scolaire et si harcèlement dans les écoles, je vous propose donc d'inclure dans ses sessions des les spécificités du cyber sexisme à caractère sexuel, incluant donc cette thématique encore trop méconnu dans la formation des polices spécialisées, je vous remercie. qu'il est dit dans le rapport que ces actions concerneront en particulier des actions de prévention contre les violences sexuelles et sexistes et le harcèlement notamment en ligne, donc pour moi c'est déjà écrit dans le rapport.

c'est favorable favorable oui merci beaucoup l'avis du gouvernement sur ces amendements, Monsieur le Ministre.

pour pouvoir à être informé du service de police et gendarmerie près de chez vous près de chez vous, près de là où vous allez, bon, c'est quand même pratique d'avoir l'adresse, numéro de téléphone le mail ses horaires d'ouverture. Pour l'instant, je crois que c'est pas très attentatoire aux libertés. 2ème sujet : est ce que vous voulez faire une pré-plainte en ligne, on peut la faire sur un ordinateur. Ben, ont proposé de pouvoir l'affaire avec une application, ce qui est, évidemment, c'est pratique. C'est pas non plus très attentatoire aux libertés 3ème sujet discuter en Direct avec un policier ou un gendarme d'ailleurs fait le moment où nous parlons, vous pouvez le faire pour me poser des questions sur le droit sur comment déposer plainte ce qu'est ce qu'il faudrait rapporter comme document ou si vous êtes une dame. Importuné dans les transports en commun et que vous êtes pas prendre le téléphone et appeler le 17. pour patienter, et puis dire bonjour, je suis harcelée par quelqu'un dans le métro ou dans le dans le bus, le pouvoir faire discrètement, comme si vous, texte à votre ami. Et en ça, je pense que c'est le renforcement de la sécurité, c'est pas le remplacement par le tout numérique du rapport à la victime, c'est un des outils qui permettent, me semble-t-il, de répondre à un certain nombre de besoins de nos concitoyens donc objectivement je, je, j'ai du mal à comprendre cet amendement 180 quant à la utilisation des robots, moi je voudrais redire avec. Le rapporteur, le rappeur, il se trouve que ce rapport il y a des moments où parfois on présente des textes au Parlement qu'on a relu et il se trouve que celui-là, je n'ai en très grande partie écrit donc je me souviens très bien, qu'effectivement je n'ai pas proposé le remplacement par les femmes et les hommes de la police nationale par des robots, mais on va le lire ensemble. Les accueil physique des brigades et des commissariats seront modernisés, c'est écrit en gras et en première ligne la brigade et le commissariat de 2032 ressembleront en rien ceux d'aujourd'hui. oui j'espère bien. Ce qui vaut en particulier pour les espaces d'accueil, c'est pas le plus top, que l'on fait des services publics, l'accueil d'un commissariat de police. Une brigade de gendarmerie, faut avouer qu'on peut faire plus riant plus accueillants. Voilà, même si c'est pas toujours des moments drôles, bien évidemment, pour tout le monde qu'on soit victime ou qu'on soit accusé ou qu'on c'est quand même toujours à un truc quand même pas super, on peut pas dire qu'aujourd'hui ce soit la plus grande humanité possible pour plein de raisons, on va pas y revenir, mais enfin, constatons-le ensemble. Un effort conséquent en terme de confidentialité d'ergonomie dans des accueils de brigades et caserne sera réalisé, je voudrais leur dire au sénateur qui a évoqué le fait qu'on devait dire les le l'intitulé de sa plainte, qu'il est un petit peu en retard de ce que nous faisons désormais si vous allez dans tous les commissariats de France, vous avez désormais devant le comptoir de la personne qui tient, c'est-à-dire un personnel civil d'ailleurs très souvent désormais le l'accueil de ce commissariat d'euros en orange et en rond bleu. C'est-à-dire que si vous êtes une femme victime de violences, vous arrivez devant le poste de du commissaire de police nationale depuis plus d'un an et désormais dans beaucoup de gendarmerie, vous ne dites même pas qui vous êtes, vous n'évoquez même pas pourquoi vous êtes là, vous n'êtes pas obligé de dire l'intitulé complet de votre plainte, ça a changé, monsieur le sénateur vous désignez l'Euro. Et notamment si vous êtes vieux victime de violence conjugale, immédiatement les services de police vous amène devant un officier de police judiciaire et cette disposition a été trouvé par des policiers de sa blessure qui, ayant compris la difficulté qu'avec certaines femmes de venir déposer plainte et d'évoquer devant tout le monde devant plusieurs personnes devant plusieurs victimes potentielles qu'ils étaient victimes de violences conjugales, par exemple, avait du mal à verbaliser les choses et c'est ce policier dans ce commissariat que j'ai rencontrés, qui a inventé ce système qu'on a généralisé, donc, désormais nous autorisons plus les policiers, a demandé l'intégralité de l'intitulé de la plainte à l'accueil, donc ceux-ci je voudrais corriger ce qui a été dit était vrai avant mais n'est plus vrai aujourd'hui. Mais au-delà des efforts nécessaires en termes immobilier, il s'agira de généraliser la prise de rendez vous en ligne. d'accentuer le déploiement des bornes d'accueil la diffusion vidéo de conduit pour optimiser les temps d'attente oui, vous êtes dans un accueil du commissariat, il vous arrive parfois d'attendre, il n'est pas anormal que des vidéos vous explique vos droits, vous êtes le que le policier par exemple tu ne peux pas vous refusez la présence d'un avocat, lorsque vous déposez plainte ou lorsque vous devez apporter un certain nombre de documents, il n'est pas, il est difficile de venir déposer plainte si on n'a pas sa pièce d'identité, peut-être qu'il vaut mieux aller chercher chez soi des choses que auxquelles on pense pas forcément lorsqu'on vient déposer plainte et qu'on est choqué dans n'importe quel service public. Et dans nos importe quel lieu public il y a parfois ses vidéos qui explique comment ça se passe dans les démarches administratives. C'est une modernité bien entendu, de même que je voudrais le dire ici ce qu'a très bien dit, le sénateur de Bresse, le robot, c'est le robot d'accueil. Qui peut tout à fait se comprendre lorsqu'on a envie d'avoir des informations par exemple, il y a plein de gens qui vont dans les services de police pour demander des choses qui n'ont rien à voir avec des enquêtes. Vous rentrez dans un commissariat pour demander votre rue, ça ça arrive tous les jours, vous rentrez dans un commissariat pour demander des copies de documents dont vous avez besoin, si vous avez envie d'ici, de déclarer la perte d'un document, une pièce d'identité, qui n'est pas allé un jour dans un commissariat pour dire j'ai perdu ma pièce d'identité, on ne l'a pas voulu, j'ai perdu et j'ai besoin de document est-ce que vous avez besoin de prendre du temps du policier pour faire cela, oui, vous pouvez le faire si vous n'avez aucune envie discuter avec une borne numérique mais vous la plupart du temps, c'est quand même beaucoup plus pratique, alors que évidemment, lorsque les choses sont plus complexes, qui demandent plus de pâte humaine, plus de travail d'enquêteur il faut maximiser le temps que nous avons de la part du policier qui peut vous accompagner, mais enfin désolé que fait la Poste. dans une poste de centre-ville, moi je trouve que dans ma mairie, je j'habitais à côté de la Poste il y a à la fois la possibilité. Pour ceux qui veulent déposer des chèques ou avoir un certain nombre de timbres, de passer par une borne numérique et puis par ailleurs, si vous avez envie de faire quelque chose de plus complexe vous allez bien évidemment voir la affaire. Son physique et il y a moins de temps d'attente et tout le monde est content, il y a un choix essai par la personne qui usagère on n'oblige personne à aller devant la borne. C'est vrai dans les mairies, c'est vrai dans la plupart des services publics et c'est vrai dans la plupart des pays qui nous entourent. Donc j'ai du mal à comprendre. Comment on peut se poser à à des choses qui me paraissent aussi aussi évidente. Non, puisqu'il serait intéressant, c'est que plus systématiquement qu'aujourd'hui la pratique, il dit : pardon pour l'anglais du mystery shopping ou de l'usager mystère sera développée, oui, parce que je suis le 1er ministre de l'Intérieur désormais à demander à des usagers mystère du service public d'aller dans les commissariats, dans les brigades de gendarmerie de me faire remonter en Direct ce qu'ils ont vu. Je le fais moi-même mais je commence à être un peu connu des services de police, alors évidemment ça ça perd un peu de sa spontanéité et il en existe encore qu'ils ne me reconnaissent pas tout à fait c'est c'est c'est donc je gagne encore un peu de temps mais plus ça avance je, anecdotes tout à fait, véritables surtout quand vous arrivez très tard le soir, sans prévenir personne, vous voyez comment vous êtes accueilli dans le service public de police ou de gendarmerie, mais bien évidemment qu'il faut pouvoir aussi contrôler la qualité de service du service public d'ailleurs, je constate que, tant sur les moteurs de recherche dis américain. public, mon service public point FR les commissariats, brigades de gendarmerie ne sont pas les plus mal notés des administrations dans leur accueil il arrive effectivement qu'on soit mal reçue, je ne dis pas le contraire, mais des efforts très importants ont été faits, donc j'ai vraiment du mal à comprendre. L'amendement 180 il me semble que c'est plutôt un renforcement du service public que ce que vous évoquez mais ainsi et dis donc un avis défavorable je donne un avis favorable à l'amendement de monsieur Bena Roche, il me semble que, effectivement, c'est légèrement redondant par rapport à ce qu'on a déjà fait adopter dans le texte mais bon voilà, comme le rapporteur des suppose pas et que le le le le thème est important, je veux évidemment donné un avis favorable à ce point, je je souhaite donner un avis défavorable à l'amendement de de madame Vogel, non pas par, par principe, mais que pour le coup, il me semble que les jeux, les choses sont très déjà très largement prévu non seulement après l'article 3 du code de procédure pénale, qui prévoit en effet de remise systématique immédiate de la copie du procès verbal de la plainte, et ça vaut pour ce sujet comme sur tous les autres, mais que par ailleurs, il nous semble qu'une très grande partie de de de cela est déjà prévu, c'est ce qu'a dit monsieur le rapporteur, et si on commence à détailler l'intégralité des sujets, ça nous paraît, ça nous paraît plus complexe maintenant j'entends bien la demande qui est faite, peut-être que je peux rappeler, Monsieur Sénateur, pour vous être agréable et parce que c'est bien normal et que c'est bien bien logique, ce que vous évoquez une nouvelle instruction aux services de police comme j'ai déjà fait précédemment, lorsque des choses correspondent pas manifestement à ce que vous évoquez, au droit, je le dis, je le dis bien volontiers Madame madame je donné un avis favorable à votre amendement, ça me paraît frappée du coin du bon sens, le qui est un grand département le plus peuplé de France. En tout cas qui envoie le plus de parlementaires à la Haute Assemblée et à Damas Assemblée évidemment mérite plusieurs maisons d'accueil pour les enfants et pour les femmes, puisque nous sommes un département malheureusement qui connaît à la fois beaucoup de population et beaucoup de violence intra-conjugales, ce serait absurde de dire qu'il en faut un par département puisque depuis la révolution, imaginer qu'un département c'est un département donc au moins je suis tout à fait d'accord avec votre votre sujet je voudrais d'ailleurs dire ici, ça vous intéressera peut-être également dans votre rapport, notamment pour les mineurs, le sujet n'est pas tant la création des maisons de protection de la famille. Que comment on traite les auditions des enfants qui sont tu, auditionné par les policiers ou par les gendarmes qui, vous le savez, des procureurs de la République demande qu'au au mot près les auditions seront retranscrites ce qui n'est pas le cas de toutes les autres auditions et lorsque vous avez un enfant de 4 5 ans qui a les mots d'un enfant de 4 5 ans qui a subi des viols. Vous avez évidemment énormément de temps, d'audition pour obtenir le maximum de caractéristiques qui pourraient aider à la suite de la procédure pénale et lorsque vous avez des policiers ou des gendarmes qui passe sept huit neuf Pour retranscrire une audition particulièrement difficile alors que, on l'a filmé et qu'on l'a enregistré, ce qui n'est pas le cas des autres auditions qui ne concerne pas les mineurs. Et que malheureusement, le procureur de la République demande au mot près la retranscription, on se dit qu'on pourrait auditionner bien plus d'enfants parce que on aurait évidemment la possibilité d'aller plus vite si on faisait des PV de synthèse et en laissant évidemment, procureur de la République, le soin de visionner les images à des moments qui l'intéresserait et écouter les bandes sonores des moments qui l'intéresserait bien évidemment pour le bien de la procédure et je pense que là, il faut qu'on avance avec les services du ministre de la justice, parce que là le le le le mieux est l'ennemi du bien et que nous nous nous perdons un certain nombre de temps et, bien sûr, on peut multiplier les maisons de protection des familles, il s'agit pas de justifier ça comme ça, mais à mon avis, d'être plus efficace devant l'augmentation des des violences sur les mineurs en comprenant les nouvelles télé. Logis l'Intelligence artificielle par exemple appliquer à ces auditions, les logiciels de retranscriptions des voix par exemple en imaginant à accepter l'idée que ces retranscriptions se fasse de manière automatique, notamment pour les pour les voix d'enfants. Me permettrez frappée du coin du bon sens pour aller plus vite dans la procédure, mais ça ne retire en rien le fait que je donne un avis favorable pour votre amendement numéro 9 l'amendement numéro 173 alors de manière extrêmement technocratique, le ministère de l'Intérieur et son état profond évoquait une comme satisfait c'est moi j'ai envie de vous dire comme si satisfait, c'est accepter, je suis bien favorable à cet amendement d'accueil dans les commissariats, brigades de gendarmerie évidemment pour les personnes à mobilité réduite, comme on dit aujourd'hui, c'est notre objectif principal, je crois que nous sommes pas l'administration la plus en retard parce qu'il y a beaucoup de gens qui vient évidemment devant les services de police et les services de gendarmerie. Sur les robots d'accueil, j'y reviendrai pas pour monsieur ben arrogent parce que j'ai défendu un avis défavorable je dois donner un ami, un avis favorable sur la même jurisprudence qu'un instant puisque c'est déjà satisfait,

sur la le caractère sexiste et sexuel dans la formation des correspondants police-sécurité de l'école ce donc madame la présidente, pour résumer nos longs débats puisque j'ai vu que vous faisiez répéter Monsieur de rapporteur je me permets donc de ne pas vous donner cette peine et de répéter moi-même un avis défavorable au 130

qui est contre qui s'abstient n'est pas adopté l'amendement 76 qui a reçu un avis défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement qui est pour.

qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté, amendement 121 avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour,

depuis 2017, le gouvernement a placé la lutte contre les violences faites aux femmes au coeur de ses priorités des progrès significatifs et indéniables ont été accomplis ces dernières années dans la lutte contre ce fléau, mais celui-ci persiste demeure et tu es surtout dans les territoires ultramarins l'enquête du CESE, menée en 2017, ou encore le rapport d'information réalisé par nos collègues Annick Billon et Michel Magras en 2020 dressé déjà ce triste constat, les violences intrafamiliales sont plus répandu en outre-mer que dans l'Hexagone, toutes les catégories sociales sont touchées par les violences physiques, sexuelles, mais aussi psychologique et économique et dans tous les espaces de vie, les traditions, les influences culturelles et religieuses peuvent rendre plus difficile pour les femmes, la possibilité d'engager des démarches judiciaires ou de quitter le coin Jogi coin juin violent l'exiguïté du territoire, conjuguée à la proximité des familles sont aussi des spécificités à ne pas négliger des moyens soient mis en oeuvre pour aider les victimes et sensibiliser les professionnels, je pense notamment à la publication, en juillet 2022 de nouveaux guides sur les violences faites aux femmes dans les Outre-mer élaboré par la Mission interministérielle Miprof à destination des professionnels ou encore à la mise en service du trente-neuf 19 joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 1 outre-mer néanmoins les efforts doivent se poursuivre et les moyens renforcés afin de lutter contre les violences intrafamiliales en outre-mer pour un accueil, une orientation et une protection des victimes plus efficace aussi au regard de nombreuses spécificités notre amendement prévoit d'apporter une attention particulière aux violences intra-famille familial outre-mer dans la formation des agents et l'accompagnement des victimes. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, on comprend tout à fait la préoccupation de l'auteur de de l'amendement et et on connaît bien la situation particulière dans les territoires d'outre-mer avec des violences intrafamiliales qui sont parfois d'une qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer en termes de violence, mais notre crainte, c'est que, en stigmatisant les territoires d'outre-mer ont oui on aboutisse à l'effet contraire de ce qu'on veut obtenir, alors que les les prescriptions qui sont données à chaque agent dans chaque territoire et spécifiquement dans les mer demande bien de prendre en compte évidemment cet aspect tout particulièrement donc moi j'aurais préféré qu'on le retire, mais un défaut je serai défavorable, non pas sur le fond mais sur l'effet contraire qui peut aboutir en stigmatisant les territoires ultramarins. je veux dire, monsieur le sénateur de Mayotte, que je comprends très bien le principe de son amendement et il a tout à fait raison de dire que parmi les augmentations très importantes de violence intra conjugales intrafamiliales les outre-mer malheureusement, ce sont les premiers en pourcentage de plaintes déposées ou de signalement à connaître ces explosions pour les raisons qui l'a évoqué lui-même et qui connaît encore mieux que moi est-ce que pour autant il faut distinguer sur le territoire de la République, un territoire où on met davantage dans l'annonce de la loi de moyens et d'objectifs que dans d'autres, il me semble pas non plus que ce soit un service à rendre surtout que les territoires ultramarins ne sont pas tous égaux, si j'ose dire dans l'augmentation de cette délinquance qui est vrai, à la Réunion à Mayotte en Martinique et et en Guyane, mais moins vrai sur d'autres territoires, notamment je pense Pacifique par exemple donc que tous les territoires ultramarins ne sont pas tous logés à la même enseigne, ce que je peux faire en donnant un avis défavorable à votre amendement sénateur c'est que vous rassurer en disant que, vu les difficultés des augmentations, on l'a vu encore très récemment, la Martinique, on a des envoyer encore plus de moyens et sans doute les les besoins en effectifs supplémentaires, notamment dans les enquêteurs spécialisés, violences conjugales, je m'engage devant vous à faire à chaque fois, comme d'ailleurs, pardon monsieur le sénateur de Brest, dans le Nord-Pas-de-Calais et en Seine-Saint-Denis, parce que souvent les la carte des violences conjugales, c'est souvent une carte de la misère, ce n'est pas exclusivement une carte de la misère, mais c'est aussi une carte de la misère de mettre davantage de moyens d'OPJ puisque dans quelques instants, j'espère, ou demain vous allez voter la possibilité promise intérieur de pouvoir affecter directement les les OPJ, donc je prends cet engagement devant vous, mais il me semble pas raisonnable de faire une discrimination dans le texte de la République. Monsieur et madame. Madame la présidente, les, les, les seuls engagements du ministre-mes détermine à retirer mon amendement, mais permettez-moi de ne pas être d'accord avec l'argument de la discrimination parce que je me suis basé notamment sur des rapports qui eux précise que, précisément, dans, dans, dans ces territoires, les violences se sont sont sont plus importantes, donc, heureusement qu'il y a ses engagements, sinon je n'allais pas retirer mes amendements juste parce que il faudrait avoir peur de stigmatiser la situation est différente et les rapports l'ont révélé, mais je, je, je, je, je m'en remets à à ses engagements et je sais qu'elles seront qui seront

Merci madame la présidente. Ces dernières années plusieurs projets ou propositions de loi visant à renforcer la lutte contre les violences conjugales intrafamiliales ou de nature sexuelle ont permis des avancées significatives, la pénalisation accrue des violences sexuelles sur mineurs de 15 ans la qualification pénale de l'inceste, la reconnaissance de l'abus d'autorité en matière d'agression sexuelle, l'allongement de la des délais de prescription ou encore l'augmentation de la portée de l'ordonnance de protection toutefois en matière de lutte contre les violences conjugales, ces progrès sont encore insuffisants dans la lutte contre les violences infligées aux femmes et aux enfants, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon édifié notamment par l'exemple espagnol l'instauration d'une juridiction spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, rassemblons juge aux affaires familiales, juge pour enfants et juge pénal est une nécessité désormais partagé tant par les associations et les différentes tendances politiques que par les principaux candidats à l'élection présidentielle, or, bien que le projet de loi annonce notamment le renforcement de la lutte contre les violences intrafamiliales cette nécessité n'est pas pris en compte, nous proposons donc par cet amendement, l'expérimentation de juridiction en charge des violences sexuelles intrafamiliales et conjugales cette juridiction sera compétente pour juger des faits de viol, d'inceste et d'agression sexuelle d'outrage sexiste et de recours à la prostitution, cette nouvelle juridiction aurait également à connaître des violences physiques, sexuelles et morales commises au sein du couple ou sur un enfant de la cellule familiale, une compétence civils la juridiction lui permettrait de prendre des décisions rapidement concernant les modalités de l'autorité parentale, du droit de visite et d'hébergement ainsi que de statuer sur l'ordonnance de protection cette expérimentation se feraient par redéploiement des moyens existants et apporterait en conséquence aux magistrats engagés pour améliorer la réponse pénale et civile vis-à-vis des violences sexuelles intrafamiliales et conjugales un levier juridique mobilisables immédiatement. Si l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. merci madame le président monsieur Ministre, chers collègues, afin de réprimer plus efficacement les violences sexuelles et sexistes, les violences conjugales et les violences intra-familiales, il est régulièrement proposé de créer, sur le modèle de l'Espagne, une juridiction spécialisée cet amendement propose d'inscrire dans le rapport annexé le principe d'une expérimentation d'une telle juridiction spécialisée avant une éventuelle généralisation s'inspirant de la démarche qui avait été retenu récemment pour les cours criminelles départementales avec mon collègue, co-rapporteur, nous ne sommes pas opposés à cette idée et à la voix de l'expérimentation ne nous paraît intéressante, néanmoins, il nous semble difficile de trancher une question aussi complexe, au détour d'un amendement à ce projet de loi sans avoir mené aucune audition aucun travail préparatoire à une telle décision en amont de cette discussion en séance publique, la seule discussion, nous avons eu, c'est la discussion que nous avons eu à 2 reprises au sein de la commission des lois et même si l'amendement n'est pas dépourvu de tout lien avec le texte puisqu'il y a évidemment un lien lié à l'outrage sexiste, vous conviendrez qu'un amendement réformant l'organisation judiciaire trouverait évidemment mieux sa place dans un texte porté dans par l'Agence plutôt porté par le ministre de l'Intérieur de plus sur le fond, de nombreuses questions restent en suspens, notamment concernant la procédure qui serait appliquée par cette juridiction spécialisée est ce qu'elle a péri compliquerait les procédures de droit commun vigueur devant le juge aux affaires familiales devant le tribunal correctionnel, devant la cour d'assises, il faut également réfléchir au Champ de compétence de cette juridiction spécialisée hôtel reconnaît tous les violences sexuelles sexuelles et sexistes plutôt au des violences conjugales et intrafamiliales, c'est une question qui est très difficile à trancher, sans avoir entendu aucun des acteurs et vous n'êtes pas sans sans ignorer que d'abord, certains professionnels expriment des réserves concernant ce projet de juridictions spécialisées et que par ailleurs, à l'instant où on se parle, le gouvernement a confié une une mission à 2 parlementaire d'abord notre collègue Dominique j'ai rien présente ce soir et la députée Émilie, sûrs de leur leur travail qui va durer 6 mois permettra d'éclairer les enjeux et de répondre aux nombreuses questions techniques et juridiques d'un tel projet c'est pourquoi madame le président, notre avis est défavorable. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui, c'est une question très importante de ce sénateur, je suis moi-même exprimé pour dire que j'étais à titre personnel mais désormais a-t-il gouvernemental puisque le 1er ministre s'est exprimé favorable à ces tribunaux spécialisés qui vont évidemment transformé le travail de la police, très certainement, je crois que le meilleur argument c'est de dire : je ne peux pas porter dans un texte de sécurité mais je pense que l'argument peut vous toucher autant de commissaires aux lois des transformations profondes du fonctionnement l'autorité judiciaire voilà ce ce serait pas, ça serait pas, à mon avis, n'y réfléchis qu'on a dit le rapporteur Hervé ni logique, donc ce n'est pas un non de principe mais vous comprenez que je ne peux pas dire hein oui sans piétiner, du coup, les compétences du garde des Sceaux.

nous ne souhaitons pas abîmé par un vote, un sujet qui, finalement, trouvent un accord assez largement partagé dans ces bancs et chez le ministre lui-même, donc nous allons retirer je ne présuppose pas que ce qui a été dit ce soir veille engagement pour la suite mais c'est c'est un sujet qui reviendra que nous porterons avec beaucoup de détermination et je crois que la cause justifie que la mission parlementaire qui est en train d'être conduite et les réflexions que nous porterons ensemble permettent d'aller au bout de cette démarche. Merci l'amendement 145 Monsieur Merci madame la présidente, par rapport à la réflexion que vous hou la la grande tirade que vous nous avez fait tout à l'heure monsieur le Ministre, je suis navré de de vous dire qu'il doit y avoir des dangereux wokistes aussi au salles votre ministère la partie relative à la jeunesse dans ce rapport fait un constat que vous avez nié tout à l'heure, mais la, la réalité est écrite noir sur blanc dans le rapport, l'image de nos forces de sécurité est aujourd'hui dégradée auprès des jeunes, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans le rapport, alors effectivement tout de suite après la raison qui a invoquée, assez, assez absurde, elle, elle nous dire, selon le rapport, c'est parce que les ex-effectifs de police ne ressemble pas assez à la jeunesse, on oublie donc les témoignages nombre de, de, de, des jeunes notamment des quartiers populaires ce sur les violences à justifier le relation peu respectueuse parfois des agents avec eux la répression violente des manifestations ou la multiplication des contrôles. Donc, nous nous trouvons que pour arriver à une telle conclusion la conclusion tout ce qui repose de de l'image de la jeune de de la police auprès des jeunes, réside dans la ressemblance entre les agents et la jeunesse, c'est une forme de déni assez extrême, mais on a bien compris qu'ici le déni était partagé sur les bancs de l'hémicycle, donc nous plutôt que de fantasmer sur une reconquête républicaine, nous pensons qu'il faut mettre la République c'est la les les principes de la République en actes notamment son principe cardinal d'égalité et donc nous proposons de nous intéresser d'abord au coeur du problème, c'est-à-dire la logement la logique parfois purement répressif dans certains quartiers, les discriminations face au contrôle la familiarité de langage, de la part des agents et une doctrine de maintien de l'ordre qui qui parle, qui permet des déviances, bref, nous proposons de prendre à bras le corps la parole de ceux qui sont au quotidien aussi parfois face aux agents et donc, nous vous proposons de sortir la tête du sable et d'affronter les problèmes en face, il faut revoir le rapport entre la que la police, entretien avec la jeunesse en profondeur, cela commence par ne pas détourner le regard, je vous remercie. Merci, merci, merci, l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. écoutez, madame la présidente, depuis le début de ce débat, nos collègues du groupe écologiste sont dans le procès d'intention dans la stigmatisation dans la volonté d'attiser les tensions dans la volonté de faire grandir les fractures, il y a un principe d'égalité dans la République, il a aussi un principe de fraternité, et là le le le texte d'orientation, il explique un certain nombre de choses sur la ressemblance, il ne nie pas la dégradation de la relation avec la jeunesse, il explique comment pourrait tenter de rapprocher de souder d'unir, de rassembler plutôt que de diviser et de toujours opposé, je suis désolé, mais je préfère le texte d'orientation du ministère que ce texte qui est un texte qui sans arrêt et discriminant et et ne désolé défavorable et fortement défavorables. Que la jeunesse de France, comme toutes les jeunesses soient rétives à l'autorité pour une partie d'entre elles, ça n'a rien d'extrêmement nouveau vous présenter ça comme si c'était la conséquence des mois et des années précédentes. Vous avez dit qu'on avait le même âge. à l'âge où nous avions le temps sans doute, d'écouter des chansons de notre temps, il y avait un certain nombre de rappeurs extrêmement connu que nous écoutons j'imagine tous, qui évoquait un peu en termes peu à même la police nationale, c'était il y a 20 ans, c'était à la fin des années c'est à la fin des années Mitterrand, c'était à la fin des années Mitterrand et je pense pas qu'on puisse dire que particulièrement technos autoritaires ni il y avait une manifestation de maintien de l'ordre qui était c'est d'autant plus vrai que les communistes participent au pouvoir, donc j'imagine, non plus que votre chaleur devait absolument parfait à ce moment-là, et donc il devait pas y avoir de difficulté particulière nos parents étaient plus jeunes, ils écoutez Renault à la fin des années 70 début des années 80 on ne peut pas dire non plus que l'intégralité du répertoire de Renaud Séchan soit extrêmement favorable à la police nationale et gendarmerie nationale même si on finit tous par embrassé un flic, finalement, hein, c'est ce que je retiens, sans doute de l'expérience par là je, mais peut-être que dans 20 ans on embrasse sous un policier quel que soit son bord politique, donc je pense qu'il ne faut pas non plus présenté monsieur le sénateur, les choses comme étant les conséquences des mois et des années précédentes, comme vous l'avez fait comme s'il s'agissait du gouvernement du président de la République qui a amené à cette situation, il y a de manière générale, une jeunesse qui peut être soit et c'était ma démonstration tout à l'heure, et elle n'est d'ailleurs pas discutable cette démonstration puisque c'est des jeunes qui sont aux militaire, c'est juste qu'ils sont policiers, c'est des jeunes qui sont gendarmes qui choisissent l'autorité, le service de la patrie, une aventure humaine et collective et puis il y a une partie de la jeunesse qui est rétive à cette autorité, bon hé ben c'est c'est normal et c'est consubstantiel au fonctionnement et c'est pas d'aujourd'hui, ça vaut depuis que l'autorité et que la jeunesse existent et cohabitent ensemble depuis donc un certain temps, donc je pense vraiment que. Ce que dire importante de Brest et et révélateur même de vos amendements, en fait, on cherche un moment favorable à la police nationale et gendarmerie en fait si on avait suivi un équilibre, on pourrait comprendre que c'est dans l'équilibre. En fait, tous vos amendements, vous êtes le seul groupe à le faire, je le constate, c'est un constat, vous êtes toujours dans le contrôle, la sanction non pas des voyous, mais des policiers. Donc c'était vrai, que c'est un un, une sorte de de démonstration à verser mais voilà je je réponds comme vous me posez la question : votre vision fait que cet inconscient des mondes sans doute le fait que, tout en disant que vous aimez la police

je dirais même si je ne suis pas du genre polémique et je crois qu'à un moment donné, il faut quand même à ce niveau-là s'exprimer parce que il faut quand même pas faire le procès permanent contre les forces de sécurité, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, y compris les sapeurs-pompiers et je crois et puis après les jeunes vous citez les jeunes mais il y a pas que les jeunes et puis il y a les quartiers urbains, il y a le monde rural et y'certes, il y a les problèmes de société, on peut le comprendre, mais de l'autre côté, je crois, on en a pas encore parlé, mais chaque, je dirais, les parlementaires que nous sommes avec les représentants de l'État dans chaque département et territoires, nous sommes associés sous l'autorité du ministre de l'Inde, monsieur le ministre de l'Intérieur, aux journées nationales, journée nationale des sapeurs-pompiers qui sont malheureusement morts en service les policiers décédés en service et les gendarmes décédés en service, je crois que ça, il faut aussi son souvenir, et ça c'est quand même le devoir de mémoire aussi, il faut le dire et et et toutes nos forces de sécurité méritent respect, reconnaissance, je vous remercie. Merci beaucoup, alors je mets aux voix donc l'amendement 145 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient n'est pas adopté l'amendement 180 et retirer l'amendement 25 madame arriver. Merci madame la présidence dont va changer un petit peu de registre, l'objectif de cet amendement et en fait de de donner corps à des une des préconisations du rapport du qui a été présenté le 21 septembre dernier prévenir la délinquance des mineurs, réalisé par 3 collègues et moi-même, cet amendement propose en fait la mise en place d'une évaluation des différentes mesures éducatives évaluation indispensable aujourd'hui en pointant que la focalisation sur les CEF nous paraît excessive, si ces centres peuvent incontestablement être efficace pour permettre une prise en charge renforcé hors du cadre pénitentiaire il nécessite une conjonction de facteurs de réussite équipe équipement articulation avec le milieu ouvert qui ça fait qu'il s'avère en fait difficile à réunir une attention plus grande doit être portée aux autres solutions proposées par la PJJ plus limité, mais parfois plus efficace et plus territorialisée et donc l'évaluation dont les critères devront être définies avec les acteurs concernés, pourrait conduire à la réorientation des moyens pour la création de nouveaux CEF vers les nombreux dispositifs existants plus pertinent. Merci beaucoup, l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Nous trouvons le le l'aspiration et la rédaction de ce cet amendement pertinente, et donc j'ai donné un avis favorable. Merci l'avis du gouvernement. Moi, je peux donner qu'un avis de sagesse parce que il me semble quand même que c'est des dispositions qui relèvent de l'évaluation des politiques publiques du garde des sceaux, mais je comprends bien le thème de votre amendement madame la sénatrice, donc à la vie de sagesse qui n'est pas contre vous, autre moment mais je ne suis pas sûr que ce soit dans un cadre du ministère de l'Intérieur, puisqu'il s'agit de gens qui purgent leur peine même centres éducatifs fermés et dans la fin de mes services, vous comprendrez, moment de sagesse. Merci, alors je mets aux voix donc l'amendement a reçu un avis favorable de la commission, un avis de sagesse du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il est donc adopté l'amendement sens monsieur Bena Roche. parlait des jeunes et que on voudrait un amendement un peu positif, nous souhaitons valoriser en fait parce que c'est une demande aussi l'engagement des jeunes nous avions déjà d'ailleurs proposé cet amendement lors de précédents textes cet amendement fait il a pas obligé de valoriser l'engagement des élèves en tant que sapeur-pompier ou que marins-pompiers en leur octroyant des points de modifications pour l'obtention des diplômes de l'enseignement secondaire, on sait tous ce que les jeunes sapeurs-pompiers constituent un vivier majeur et indispensable pour le volontariat, il nous semble pertinent de récompenser les cabinets, les cas les qualités humaines des jeunes volontaires en n'impactant leur parcours scolaire par des points de bonification lors des examens nationaux comme le brevet ou le bac, comme tout à l'heure d'ailleurs je ne suis pas revenue, monsieur le rapporteur, que. Malgré que le midi était prêt à accepter qu'une expérimentation qui marche fasse partie de sa programmation pour les 5 ans à venir, parce qu'il estime qu'elle devra être développé ou donner un avis défavorable sur les LGBT plus en accueil au commissariat, j'ai toujours pas compris,

pour ces jeunes là dans un plan d'orientation et de programmation ministérielle qui pourra aller plus loin dans les 5 ans à venir, il est destiné à à cela, donc j'ai 2 comprendrait pas là encore à la vie où le gouvernement annonce une campagne de recrutement des pompiers volontaires sur donc très importante, pompier volontaire, j'en ai discuté et avec le Grégory Allione et avec le contre-amiral des des marins-pompiers, à Marseille, je veux dire c'est quelque chose qui fait partie de leur façon de concevoir la possibilité d'arriver aux objectifs que vous avez vous-même déterminé avec une campagne de communication, mais qu'il faut accompagner avec des initiatives complémentaires s'en études c'est pas moins intéressant que la musique ou qu'une autre option qui permet d'avoir un peu de poids, donc voilà. Si cher collègue, l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. un amendement de quasi identique en disant bien sûr qu'il faut voir le valoriser l'engagement des jeunes sapeurs-pompiers mais qu'il ne faut pas introduire par ce dispositif, une distorsion à l'égard des jeunes qui exerce d'autres activités bénévoles en août, le principe d'une bonification va à l'encontre du caractère désintéressé de l'engagement comme jeune sapeur-pompier donc défavorable pour les mêmes raisons, qu'on l'avait dit du temps de la loi Matra. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui, et j'ajouterai, par ailleurs, Monsieur le Sénateur, que ce que votre moment il prévoit finalement d'aider pour les les diplômes secondaires dont le bac si je vois bien votre démonstration, c'est quand même assez difficile à organiser, en revanche, le gouvernement a déjà prévu que pour les jeunes sapeurs-pompiers, ils peuvent rentrer ces modifications pour Parcoursup. Et donc c'est une me semble-t-il chose de très de très positif, donc je me rangerai à la vie de monsieur le rapporteur, considérant qu'une grande partie déjà de votre demande est exaucé de reconnaissance. Merci, alors je mets aux voix l'amendement sens qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté à mon nom 79 Monsieur Bénard Roche. Alors on va revenir sur un sujet qui va, qui un peu fâché, donc je m'en excuse puisque les positifs marche pas bon en fait, selon la commission consultative des droits de l'homme, les forces de l'ordre à te pouvoir d'appréciation extrêmement étendue. Sur l'opportunité de contrôler ou non une personne, le défenseur des droits, reconnaissez que l'enchaînement systématique des contrôles d'identité revenait à généraliser dans certaines zones du territoire des pratiques de contrôle d'identité discrétionnaire, ça, c'est pas des gauchistes vos qui se qui vous parle, c'est la commission consultative des droits de l'homme, c'est le défenseur des droits, les contrôles d'identité abusifs ou discriminatoires sont une réalité quotidienne pour bon nombre de personnes en France, le contrôle au faciès, excusez-moi du terme fait quand même individu peut être contrôlé trois ou quatre fois dans la même semaine, cette pratique a pour effet clair de générer des tensions entre les forces de l'ordre et la population, la Cour de cassation, pas des veaux qui gauchiste, le 9 novembre 2016 avait rappelé que contrôle d'identité fondée sur des caractéristiques physiques, associé à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable et discriminatoire, il s'agit d'une faute lourde qui engage la responsabilité de l'État, le Conseil constitutionnel avait rappelé également que la pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires discrétionnaire est incompatible avec le respect de la liberté individuelle, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, ainsi que le défenseur des droits recommande pour lutter contre ces pratiques abusives, la mise en place d'un système de traçabilité des contrôles d'identité, par le biais de la remise de récépissé à l'usager après chaque contrôle d'identité, cette mesure. Défendue aussi par des associations depuis plusieurs années, si elle ne constitue pas la solution miracle pour lutter contre les discriminations est un moyen pour limiter la latitude important dans la sélection des personnes interpellées si la formulation de l'amendement ne vous convient pas, nous le comprenons, mais ce rapport annexé est une feuille de route pour les prochaines allez il paraît plus que temps d'y intégrer une réflexion sur les conditions et dérives des contrôles qui en prison qui empoisonne la vie de certains, je termine rarement dans le 16ème arrondissement.

que il y a eu longues explications de des rapporteurs du ministre, et cetera et qu'on n'a pas changé tous les modalités de réalisation des contrôles d'identité sont précisés de manière limitative et respectueuse des droits de l'homme par la 78 2 du code de procédure pénale et il y a pas de contrôle dit de d'identité à l'initiative, ou des choses de ce type, je suis désolée, moi je suis le ministre du logement qui a imposé aux agents immobiliers, la charte de non-discrimination dans l'accès au logement, pour des raisons de faciès, donc je sais de quoi je parle, et franchement je trouve que vous poussez le bouchon très loin : avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre, même avis. Merci, je mets aux voix donc l'amendement 79 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement ah Monsieur Bénard Roche, pardon, excusez-moi.

tout à fait légitime la mienne l'est tout autant, celle de la Cour de cassation, celle du de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, celle de la défenseure des droits, celle du Conseil Constit. Fusionnel me paraissent aussi digne d'être écouté, donc on peut pas rejeter comme ça d'un revers de main sous-réseau de prétexte quelconque, J'ai pas terminé, je suis désolé, ça ne fait pas de minutes, bon c'est peut-être vous, mais il y a des gens qui écoutent, ils en ont pas assez je terminerai en disant que, par exemple, il a été notoirement vérifier et et a annoncé y compris dernièrement dans les derniers chiffres été donné qu'il y a une disparité énorme par exemple dans les contrôles concernant les attestations Covid. En fonction des endroits où elles avaient lieu et chacun d'entre nous a pu le constater et ça nuit à l'efficacité du travail d'enquête et de poursuites pénales, ça, ça le nuit ça nuit aussi à la confiance entre les citoyens et la police, voilà c'est tout. Merci Madame Lienemann. puisque depuis plusieurs années, on voit que des tensions et une incompréhension peut s'opérer entre une partie de la population jeune ou pas jeune d'ailleurs, et nos forces de l'ordre et pendant des années on nous a expliqué, pour être sûr que cette incompréhension qui moi je l'ai observé dans certains cas minoritaires certes, mais dans certains cas, on a quand même le sentiment d'un acharnement qui peut d'ailleurs naître d'une certaine difficulté pour les forces de l'ordre appréhender les problèmes auxquels doit faire face, alors pendant un moment, nous à dire les caméras embarquées là qui vont permettent de donner des garanties, j'observe qu'on n'a pas atteint le seuil de confiance réciproque qui est nécessaire dans une république entre les entre les citoyens et les forces de l'ordre dans certains territoires et dans certains cas, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre en oeuvre des processus qui habitent qui qui sont pas de nature enlever l'autorité aux forces de police, à partir du moment elles sont généralisés et que ça devient une pratique reconnue, on verra d'ailleurs que, dans certains cas, les gens ex-exagère parce qu'il y a pas autant de contrôle qu'on le dit mais je ne vois pas en quoi cette transparence est de nature à affaiblir la relation entre la police et la population, ni même l'autorité de la police. Merci, monsieur le Ministre. Merci. Il y avait un présente, je suis toujours frappé par ce débat puisque. On ne parle pas de chose qui. Correspondent à la réalité du droit. Non, la Ministre, pardon, j'ai beaucoup de respect pour votre engagement, mais vous avez, vous avez dit une bêtise juridique, ce ne sont pas les policiers et les gendarmes qui font d'initiative des contrôles d'identité.

soit parce que le procureur de la République donne des réquisitions de transiter dans des lieux particulièrement criminogène. Par exemple, les gares. Non mais c'est le procureur de la République, c'est une politique pénale, vous m'avez demande de la réforme de la police nationale, tous s'expliquer qu'il fallait respecter l'indépendance de la justice ne pas commenter les instructions des procureurs de la République et des magistrats et ne pas remettre en cause l'indépendance de la justice parce que on a eu ce débat pendant 2 heures, là je vous dis que quand les policiers et les gendarmes contrôlent pas autour des gares ou dans les stations de métro, c'est qu'ils ont des réquisitions du procureur de la République, très bien mais soit la justice est indépendante, soit elle l'est pas quand elle donne des instructions pour dire aux policiers dans ce périmètre là vous pouvez contrôler, excusez-moi, il y a pas vérité ici et et ne pas vérité là quand ça vous arrange, selon les services de police, les policiers et gendarmes, il contrôle quand ils ont des réquisitions de contrôle voilà, après il y a un 2ème cas où ils peuvent contrôler l'identité d'une personne. C'est lorsqu'ils sont officiers de police judiciaire. C'est quand même assez peu évident dans la vie de tous les jours, ça peut arriver, y compris dans les effectifs de bac, il a des OPJ dans les effets de de bac à partout et cette OPJ lorsqu'ils ne respectent pas la déontologie et des règles du contrôle, le procureur de la République, il retire son habilitation, ça arrive très souvent, voilà que le procureur exerce d'opportunités un contrôle. Puisque ce n'est pas moi qui donne le PJ c'est le procureur de la République qui donne cette OBJ après un examen d'ailleurs réussi, présidée par un magistrat et la 3ème situation pour lesquelles un policier d'initiative fait un contrôle, c'est lorsqu'ils constatent une infraction un Crime ou un délit. Quelqu'un viendrait à dire sortie du Palais du Luxembourg, on a tué, on m'a volé mon sac, le policier bien sûr après ces actes sont d'ailleurs contrôlé par le les juges du du viendra dire bon ben voilà, j'espère quelques construire pour s'apercevoir si c'est bien cette personne qui a été vu en train de voler le sac de madame, monsieur, monsieur. Mais il n'existe pas, Madame la Ministre, Monsieur le Sénateur, dans la loi française la possibilité pour les policiers et pour les gendarmes de faire des contrôles d'identité, d'initiative, si vous pensez que ces contrôles d'identité sont trop nombreux pour les raisons que vous évoquez, il faut l'évoquer lorsque la politique pénale est prise soit dans un débat politique pénale puisque c'est vous qui l'avait autorisé par la loi de la République soit expliqué qu'une partie des procureurs de la République sont donc manifestement organisée pour c'est pas ce que vous avez dit Madame la Ministre, parce que tout ce que vous avez dit monsieur le sénateur pour répéter un certain nombre de contrôles. Pour des personnes en raison de leur faciès est-ce que vous avez dit ça veut donc dire que les procureurs de la République organise un contrôle raciale au faciès, je sais pas comment vous l'expliquez, en France, donc ce ne sont pas les services de. Police qui le font, ils le font toujours, sous l'autorité d'un magistrat, mais, Monsieur le Sénateur, auriez-vous la même démonstration lorsque je vous dis que la plupart des contrôles fiscaux sont faits pour les personnes qui touchent le plus d'argent. Mais c'est exactement la même démonstration, ceux qui sont le plus responsables de fraude fiscale sont en proportion, les gens qui gagnent plus d'argent je suis très sérieux parce que dans ce débat que j'ai tenus ici sur la fraude fiscale, vous m'avez interpellé, pas vous mais votre groupe pour me dire mais il faut accentuer l'homme de contrôles fiscaux, chez qui, ben on peut se poser la question puisque ils ont plus d'argent, par l'absurde que vous évoquez, elles démontrent vos propres arguments, la vérité c'est que vous ne faites pas confiance aux forces de l'ordre, la vérité c'est que pour vous, la parole de la personne contrôlée vaut la personne du contrôleur, la vérité c'est que pour vous, un homme en uniforme, une femme en uniforme et par nature suspect la vérité, c'est pas des jeunes qui n'est pas l'autorité, c'est votre groupe politique.

on va, on va quand même reciter la commission consultative des droits de l'homme qui dit que les forces de l'ordre ou un pouvoir d'appréciation extrêmement étendu sur l'opportunité de contrôler ou non une personne c'est pas moi qui le dis, c'est elle, elle dit aussi dans son avis sur le rapport entre police et population visant à rétablir la confiance entre la police et la population que les jeunes policiers en fonction de certains quartiers dits sensibles, témoigne d'un manque d'encadrement par des policiers plus senior n'étant pas originaire par exemple d'Île-de-France ne souhaitant pas y rester et pouvant mener à des actions de type contrôle au faciès, le rapport de la Cour des comptes de décembre 2019 soulignent notamment en ce qui concerne Paris, que la préfecture de police souffrent d'une faible attractivité d'un déficit en personnel, confirmé et d'un grave sous-encadrement cet amendement, cette fois-ci, vise à aider nos forces de l'ordre vise donc à renforcer l'encadrement des jeunes policiers dans les quartiers dits sensibles, par des policiers plus seniors seniors en augmentant l'attractivité de ces zones afin de réduire le mal-être policier. Merci et puis la commission, monsieur le rapporteur défavorable, monsieur le Ministre, de l'avis du gouvernement, même avis je mets aux voix donc l'amendement 129 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour, qui est contraint qui s'abstient n'est pas s'adopté l'amendement 88 monsieur Bena Roche.

on est accusé, nous en les citant d'être des extrémistes gauchistes et 9 excités en fait un certain nombre de choses et qu'essayer de résoudre des situations, donc je vais, je vais prendre que deux minutes je prendrai ensuite le reste en fait, cet amendement il est aspiré à la fois des travaux d'une association qui s'appelle Acer action sécurité éthique républicaine et d'une proposition de loi d'ailleurs de nos collègues députés qui s'appelle François Ruffin. Oui, ça c'est pas un bon point pour moi je sais et il rejoint donc le ministère de l'Intérieur a renoncé aux pratiques d'immobilisation l'étal qui ont conduit à de nombreux accidents mortels, je peux vous en citer quelques-uns, Cédric vaches ou via qui est décédé le 5 janvier 2020 après une interpellation suite à une fracture du larynx provoquée par une clé d'étranglement à Mathias au sol 16 novembre 2017 condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour la mort de Mohamed Boukrourou pour traitement inhumain et dégradant, suite à son interpellation immobilisation 19 juin 2018 Cour européenne des droits de l'homme, de nouveau, reconnaît la responsabilité de la France pour négligence dans le décès d'Ali Ziri dans la mort découleraient de pliage ventral. 2007, sûrement un peu plus haut à la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour le c'est Mohamed Saïd, qui avait été maintenu au sol pendant 35 minutes dans une position susceptible d'entraîner la mort par asphyxie qui était en forme d'immobilisation hautement dangereuse, très ont d'ailleurs le directeur général de la police nationale, Frédéric Veaux a entériné, dans une note de service, le renoncement à toute occasion de la tactique de clé d'étranglement et de celui de plaquage ventral le plaquage au sol est également une tactique policière controversée ayant provoqué au moins 4 cas mortels en France depuis 2005 qui est interdit en Suisse, en Belgique, dans certaines villes des États-Unis, alors qu'il reste toujours autorisées et pratiquées en France. Si certaines de ces pratiques sont déjà est prohibé par la direction générale de la police nationale via des notes destructions, elles ont encore été parfois pratiqué sur le terrain. Merci, c'est bien l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. J'ai dit que systématiquement, quand on serait sur le Champ de travail d'une mission d'information, ce qui est le cas. On attendrait les conclusions de cette mission après les auditions donc Madame Carrère et Madame Di Folco son rapporteur d'une mission sur les moyens d'action, les méthodes d'intervention de la police et la gendarmerie, j'ai donc donné un avis défavorable à tous les amendements qui traite de cette mission dans l'attente des conclusions de la mission. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre, ma ma vie merci donc je mets aux voilà monsieur Bena Roche. Par l'explication de vote, donc du coup du bien sûr je je comprends ce qu'a dit le le rapporteur, c'est quand même une précision a demandé au midi parce que c'est quand même une une loi de programmation et d'orientation, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait mettre des trucs sur la police judiciaire en attendant que la mission ait lieu, parce que de toute façon on pouvait quand même le mettre, donc je pense que parcourir en 100 pour 100 pour émettre des trucs là dessus, quand même, en attendant la mission parce que de toute façon après la mission, on fera le nécessaire en fait ça, ça me paraît cohérent alors si certaines de ces pratiques sont déjà prohibé par la direction générale gelé. Le groupe écologiste lui demandent leur prohibition formelle par le ministère de l'intérieur par une inscription dans la loi, nous espérons juste pour l'instant une clarification à venir de la doctrine du ministère de l'Intérieur, si les techniques d'immobilisation sont un outil nécessaire des forces de l'ordre reste que leurs conséquences potentielles doivent être prises en Côte dans leur mise en oeuvre, ça pourrait être une bonne orientation du ministère de l'Intérieur, il reste dommage de ne pas vouloir interdire les plus dangereuses pour pour faire l'économie d'une formation initiale, plus complète et plus complexe, l'économie d'une formation continue plus adapté et plus fréquentes. Merci, alors je m'envoie l'amendement 88 qui avait reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient ne pas adopté 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 82 monsieur Bena Roche. Alors, cet amendement est inspirée de la proposition de loi qui avait été déposée ici-même et défendu de notre collègue sénatrice à l'époque député actuellement, Sophie Taillé-Polian, qui visait à rétablir la confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre en demandant au gouvernement la création d'une autorité indépendante, rattachée au défenseur des droites des droits, pardon, en charge de la déontologie des forces de l'ordre, les instances actuelles chargée d'enquêter sur les bavures policières, l'IGPN pardon ne remplissent pas leur rôle, défaut de célérité des enquêtes manque d'impartialité, manque de transparence, le défenseur des droits, le répète depuis de nombreuses années, le respect de la déontologie par les forces de l'Ordre constitue un élément central de la confiance des citoyens à l'égard des institutions, d'ailleurs, ça paraît évident pour tout le monde en 2019 les réclamations contre la déontologie des forces de l'ordre ont augmenté de 29 la police des polices, s'est vu confier 1460 enquête judiciaire, la même année dans plus de la moité des accusations de violences des forces de l'ordre, le défenseur des droits a également demandé l'engagement de poursuites disciplinaires d'autres anti-dossiers aucune de ces demandes été suivies d'effet, quant aux sanctions pour discrimination, elles sont, selon la CNDH Cncdh quasi inexistante, le président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé la création de n'organe de contrôle parlementaire des forces de l'ordre au au retour en Corée défini lors d'un discours à l'école de police de Roubaix le 14 septembre 2021, cette annonce n'a pas été suivies d'effet, notre groupe propose donc au gouvernement d'inscrire ce projet directement dans sa programmation, la réforme d'ampleur de l'IGPN annoncé par le précédent ministre de l'Intérieur, le 8 juin 2020, sobre, selon les mots du professeur de droit Olivier Kahn avoir rejoint le vaste cimetière des promesses de circonstance destinée à apaiser l'opinion publique après une bavure l'État toc doit de toute urgence, réformer la culture policière, ce qui suppose aussi de modifier cette. Cette loi, cette appréciation des bavures policières. Merci, si le l'amendement 121 messieurs dur. Merci madame la présidente, premier deux trois amendements qui s'inscrivent dans une réflexion assez large sur les relations entre la police et la population, le paragraphe de 2,7 du rapport annexé s'intitule garantir la transparence et l'exemplarité de l'action des forces de l'ordre, il souligne à juste titre, que la demande sociale d'exemplarité dans le comportement des forces de sécurité s'accroît et s'exprime à travers une revendication d'indépendance et de transparence et de la manière dont celles-ci sont contrôlés, c'est des sujets que nous avons évidemment abordé au bout de la sécurité qui qui font l'actualité, malheureusement, il me semble que les pistes qui sont envisagées par le ministère, d'en prendre pas cette direction, même si nous prenons acte de la création d'un comité d'éthique auprès du ministère de l'Intérieur et de la modernisation annoncée des plateformes de signalement effectué auprès des inspections générales alors le rapport annexé à raison de rappeler que les mécanismes actuels de contrôle interne des forces de l'ordre sont obligés de récurrents de critiques récurrentes justifiée en raison de leur manque d'indépendance qui entretient un soupçon de partialité et ne favorise pas toujours l'amélioration des relations entre la population et les forces de sécurité, nous en connaissons la raison, outre l'effet de corps à la composition actuelle des organes de contrôle qui comprennent majoritairement des policiers, des gendarmes, ces derniers sont rachetés rattachée organiquement au ministère de l'Intérieur, via la direction générale de la police et la gendarmerie de ce fait, il y a une forme d'entre soit professionnel qui entretient une culture qu'on pourrait dire, le corporatiste, alors il nous semble, au travers des propositions que nous formulons qu'on pourrait s'inspirer de ce qui nous a été finalement proposées au sein du Beauvau de la sécurité, l'exemple emblématique de officie britannique qui est un office indépendant du comportement policier qui est chargée d'instruire les affaires les plus graves qui peut s'autosaisir qui ne rend pas compte à l'exécutif, qui dispose de son propre budget de ses propres enquêteurs qui ne sont pas rattachés au service actif de la police et dont les directeurs ne peuvent pas du fait de la loi, être des policiers le critère d'indépendance du contrôle de l'usage de la violence par la police est essentiel dans un état de droit et la condition de tout en légitimité dont les autorités qui contrôlent collègue n'aurait jamais dû se démarque. Alors l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Ce que les auteurs de ces deux amendements ne mentionne pas, c'est qu'une réforme des inspections, a d'ores et déjà été lancée pour rendre plus lisible leur travail et plus efficace leur efficacité. pour renforcer leur efficacité. Par exemple, dans ce rapport il est prévu la publication des rapports des inspections pour la transparence, le renforcement de la formation matière de déontologie des policiers et gendarmes ou encore l'instauration au sein de l'inspection générale de la police nationale, d'un comité d'évaluation de de la déontologie, incluant des représentants de la société civile avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement, monsieur le ministre. C'est une question très importante, qui évoque le sénateur durera et bien sûr ce que vous avez évoqué, monsieur le sénateur encore un amendement de confiance vis-à-vis des forces de l'or par définition même si sénateur torture à temporiser, si j'ose dire, votre élan dans votre folie de contrôle et de sanction, une sorte de d'autoritarisme qui qui ne vous ressemble pas sur les autres sujets que nous abordons, mais je veux bien avouer que les questions des inspections, ils ont plus intéressant à évoquer ici que nous n'avons pas de faits divers particulier dans l'actualité et nous permet d'avoir des discussions. Au moins. C'est jamais évident lorsqu'un fait divers, très important, est arrivé, d'abord je me permettrai de vous faire remarquer, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'il y a paradoxe dans nos discussions sénatoriale. Que font les magistrats instructeurs. Ils saisissent dans leur libre choix, article 12 du code de procédure pénale, le service instructeur qui va enquêter. Et c'est donc tout à fait libre. Que le juge d'instruction, procureur de la République, choisi de saisir ou pas, l'IGPN ou du GIGN ou n'importe quel autre service de police ou de la porte culotte service de gendarmerie. Donc l'IGPN sont avant tout un service enquêteur. De la police, je mets des guillemets judiciaire d'enquête qui répondent non pas une auto-saisi les bien saisi de magistrats et, comme nous venons de répéter que nous sommes tous très attachés à la liberté de choix. Des services du par le magistrat instructeur, là encore, je me permets de dire que c'est sa liberté très grande de saisir l'IGPN ou de ses alliés GIGN et que si c'était une un service d'enquête qui n'étaient pas conformes aux règles déontologiques à la démocratie et l'accueil de l'état de droit et un autre, soit il ne saisirait pas ses services. Première paradoxe par rapport aux discussions du début de notre discussion sénatoriale 2ème paradoxe votre intervention, monsieur sénateur et juste, mais si je peux me permettre et les dater. J'ai depuis le Beauvau fait de nomination. Qui n'ont pas de précédent dans l'histoire du ministère de l'Intérieur. J'ai nommé un magistrat. à l'inspection générale de gendarmerie nationale et j'ai nommé une magistrate judiciaire qui plus est, procureur de la République à la tête de l'IGPN. C'est la première fois que le ministre de l'Intérieur propose non pas des policiers, non pas des gendarmes n'ont pas des préfets, non pas des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, mais des magistrats. De leur judiciaire pour pouvoir être effectivement chef d'enquête ou directeur, on en reparlera d'administration sur ces 2 postes,

Donc, il est désormais faux de dire que ce soient des policiers ou des gendarmes qui dirige ces inspections. Troisièmement. Aujourd'hui l'IGPN et l'IGGN ne sont pas simplement des services d'enquête sur ce que fait mal ou ce que ferait mal les policiers et les gendarmes, c'est aussi un service d'inspection à la main, si j'ose dire, du directeur général ou du ministre de l'Intérieur, comme il y a une inspection générale des affaires judiciaires, comme il l'Inspection générale des finances, comme il y a une inspection générale de l'environnement. C'est donc mon inspection, si j'ose dire, en tant que ministre-qui me rend des rapports d'ailleurs personne n'a contesté le fait que l'IGPN était qualifiés pour on ne rapport sur la réforme de la police judiciaire, donc vous pourriez au moins dans vos un moment si je peux me permettre distinguer la fonction enquêtrice de la fonction d'audits inspection il n'appartient à personne, ici, de se dire : tiens, les services d'inspection de la nuit, ça la justice devrait être indépendant ou l'IGF devrait être indépendant de Bercy, parce qu'ils sont jugés partie c'est le principe, ce serait une révolution ce c'est, c'est le principe des services d'inspection que dépendre de son ministre de ces directeurs généraux, c'est bien le même et vous savez les l'IGPN et Gégé ne sont pas les seuls à pour être saisis par la justice, l'IGF. Alors c'est vrai que c'est moins courant mai et parfois saisis par la justice pour faire des contrôles, notamment parce que le secret fiscal par exemple a été dévoyé et personne ne vient à dire : ben non, ils se jugent entre eux. Il y avait un certain nombre effectivement de difficultés dans les fonctionnements de l'IGPN et gégène, à commencer par le faible nombre d'enquêteurs que nous avons renforcé, à commencer par le fait que on ne jamais les rapports, monsieur le rapporteur a eu raison de souligner que j'ai désormais décidé de les publier sur tous publics, à commencer par le fait que les directeurs généraux, quand il avait les rapports ne prenait pas toujours les sanctions, en tout cas il pas encadré dans le temps, j'ai désormais dit en moins de 2 mois le DGPN ou DGGN doivent prendre des sanctions qui correspondent à la demande IGPN et l'IGGN, donc ces améliorations ont été très largement souligné par tout ce que vous avez cités et, notamment, la défenseure des droits que je remercie pour cette remarque notamment le fait qu'on ait mis des magistrats à la tête de ces inspections. Alors je terminerai par dire quand même que c'est une drôle de critiques que dire vous n'avez pas créé le l'organe de contrôle parlementaire bah oui a séparation des pouvoirs, que les chambres crée l'organe de contrôle parlementaire c'est c'est pas le l'exécutif qui peut intervenir dans le fonctionnement du Sénat où l'Assemblée nationale est changé son règlement, il vous appartient. Nous avons dit nous, que nous étions absolument favorable à ce qu'un organe parlementaire qui contrôle dans chacune des chambres de l'action du Parlement comme il a cru que l'action de des forces de dedans, il contrôle l'action des services de renseignement donc Monsieur le Sénateur, j'imagine que cette interpellation ne s'adressait pas à l'exécutif, mais plutôt à votre assemblée et puis enfin, je dirais que si il y a bien des choses qui sont intéressantes dans les épreuves cinématographique nous vivons, c'est que chacun a pu constater que l'IGPN n'était pas la reproduction du corps d'ailleurs les policiers et les gendarmes, en général on image assez peu positif de leurs inspections. Pour ceux qui ont vu Bac Nord nous y voyons sans doute une image de l'IGPN qui n'est pas à l'honneur, sans doute le le la police nationale dans la mesure où on a l'impression que ces policiers ont été broyées par un service d'inspection technocratique venant de Paris par les boeuf tels qu'on les appelle dans la police et ça nous fait plaisir absolument à aucun policier de réponde de ses actes devant l'IGPN et l'IGGN et c'est pas une partie de plaisir, bien évidemment, parce que c'est un vrai service enquêteur, vous savez bien, ils ont une haute conscience de leur travail d'enquêteur alors après il y a un débat de société, moi je veux bien l'avouer que ce débat existe avec Monsieur dur est ce qu'on doit imaginer d'autorité initiative indépendante faut-il une nouvelle fois que le pouvoir exécutif se dessaisissent de son pouvoir pour pouvoir effectuer disciplinaire dans son ministère. Mais moi, je, je n'ai rien que les autorités illustrative indépendante vous renier, de plus en plus le pouvoir de l'exécutif et du législatif, vous n'aurez pas ce débat avec une autorité d'initiative indépendante, monsieur le sénateur, ce qui est sûr, c'est que vous ne pourrez pas à le président la président de l'Autorité initiative indépendant Lucic pour répondre à à vos interpellations à vos critiques et à ces échanges, réfléchissons bien avant de donner de nouveaux à pouvoir la démocratie britannique a aussi ses défauts, et je ne suis pas sûr que toutes ces qualités sont transposables dans notre démocratie. Deuxièmement, faut-il distinguer le service d'enquête du service de conseil et d'audit, je ne le crois pas, non plus, on peut avoir ce débat bien évidemment entre nous parce que des erreurs factuelles que nous voyons faites par telle ou telle personne, on en tire des conclusions bien sûr sur la personne et la sanction qu'elle doit avoir, mais aussi sur la chaîne qui a malheureusement cette personne à faire ce genre de fautes, notamment le manque de formation, notamment le manque de matériel, notamment le manque d'ordre clair de la part des services hiérarchique ne croyons pas que quand on prend une sanction contre un policier qui a fait une bêtise ou qu'il a commis un délit, nous ne posons pas des questions également à l'administration elle-même et on essaie de changer un certain nombre de process, quand on fait son travail sérieusement si vous distinguer de service d'enquête du service, comment dirais-je d'audits et de conseils, vous ne permettrait pas, je crois, la plus grande fluidité qui relevé, je voudrais aussi vous soulignez que la défenseure des droits qui est déjà une autorité administrative indépendante elles-mêmes et de saisie de manquements sans passer par l'IGPN par GIGN de ce que pourrait faire des fonctionnaires de police qu'elle existe déjà en très grande partie elle même contrôle l'action de l'IGPN et l'IGGN, par l'intermédiaire des rapports d'ailleurs à leurs débuts en en témoigner. Monsieur le rapporteur dans le tables rondes le boulot de la sécurité parce que même le défenseur des droits étaient étaient présentes, alors évidemment, comme toute inspection comme tout service d'enquête tout n'est pas absolument parfait, bien évidemment, vous avez raison, mais je crois que les améliorations successives qui ont été déposés et les réformes que nous avons pu faire en y mettant des magistrats à la dette, en publiant les rapports en prenant les sanctions sous 2 mois, en nous inspirant de des bonnes pratiques, tout en considérant que il n'y a qu'au ministre de l'Intérieur, qu'on demande de se séparer son inspection quand tous les autres ministres peuvent garder l'inspection ne me paraît pas très cohérent, donc ce sera un avis défavorable pour l'amendement du groupe écologique, je veux dire du même principe qui dépose évidemment sa transformation des inspections, c'est un avis défavorable pour Monsieur pour des raisons je crois très argumenté que j'ai pu lui opposer laissons aussi le temps, monsieur le rapporteur, de voir ce que tu changeras comme pratique et comme organisation le fait qu'on ait mis des magistrats à la tête de ces inspections, avouez que ça fait seulement quelques mois et que ça mérite sans doute un peu de temps, surtout que vous savez bien que c'est une révolution pour la maison. Merci, alors je vais mettre aux voix l'amendement 82 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté, amendement 121 avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient n'est pas adopté

et du meilleur encadrement des interventions de police n'est pas du tout abordée au fond pourtant, la multiplication des tensions et des incidents parfois graves entre les forces de l'ordre et les participants aux manifestations auraient dû conduire le ministère à s'interroger sur les conséquences de la doctrine modifié du maintien de l'ordre et de sa mise en oeuvre, cette dernière a apporté des garanties mais prévoit le durcissement des conditions du maintien de l'ordre dans la, dans une logique de confrontation pouvant aboutir à de très fortes tensions au contraire la relation entre la police et la population ne va être fondée sur une recherche de confiance en privilégiant le contact avec la population, ce constat fait partie d'une logique d'ensemble que nous avons dénoncé représentant l'amendement numéro 21 contre risque de réintroduire la politique du chiffre cette logique conduit à évaluer les agents de forces de sécurité non dans leur rapport étroit et la bonne connaissance de la foule qu'il côtoie, mais parce qu'ils atteignent par exemple un certain nombre d'interpellations, il serait nécessaire de recentrer le maintien de l'ordre sur sa mission de prévention et d'accompagnement des manifestations, le choix du modèle dit de désescalade permettrait de diminuer la conflictualité, cela suppose que les services de renseignement soit connaisseur des profils et des motifs au coeur de la contestation cette orientation suppose de développer le dialogue et la concertation, condition d'un rapprochement dans les relations police-population de réexaminer avec courage, l'équipement, des policiers, des gendarmes intégrée aux stratégies du maintien de l'ordre et enfin de renforcer la formation initiale et la formation continue des forces de sécurité, je vous remercie. si l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure sur cet amendement, le suivant et d'autres qui vont suivre, je vais donner un avis défavorable puisque. Ils sont complètement dans le Champ de la mission d'information sur les moyens d'action et méthodes d'intervention de la police et de la gendarmerie dont Madame Carrère Madame Di Folco, ce sont les rapporteurs défavorables. Merci, monsieur le Ministre, de l'avis du gouvernement. très très rapidement, j'ai moi-même évoqué une crise d'ordre public, je ne veux pas mépriser votre intervention, monsieur le sénateur, vous avez raison, en partie, il faut améliorer la formation, c'est ce que j'ai dit : on a passé de 12 mois de 8 mois 12 mois la formation initiale et on recrute 705 formateurs pour la formation continue, il faut améliorer le matériel vous avez raison, je ne partage pas tout à fait l'opinion que la désescalade se fait que par le matériel, il y a des moments où il n'est pas nécessaire que les policiers ou les gendarmes du maintien de l'ordre et un matériel lourd, vous avez tout à fait raison ça peut créer quelque chose, non positif et aller vers l'escalade, comme vous l'avez dit, il y a des moments où ça se justifie donc je pense qu'on on pourra en discuter évidemment, vous savez, on n'est pas du genre à demander toujours le matériel lourd parce que le principe des mobiles, c'est qu'ils soient mobiles, plus c'est lourd, moi c'est facile pour bouger donc indépendamment de l'aspect philosophique et l'aspect pratique et je peux le partager, je voudrais vous dire quand même que le meilleur moyen d'améliorer le maintien de l'ordre, il y a le schéma du maintien de l'eau pour la première fois, nous l'avons écrit, il a été retoqué par le Conseil d'État, je l'ai réécrit et d'ailleurs il a été validé par la profession, j'aimais évidemment des guillemets, parce que c'est plus complexe que ça, notamment de ce qu'il a présenté les les journalistes puisqu'on a fait énormément d'avancées même si tout n'est pas absolument parfait une science très difficile que celle du maintien de l'ordre, je voudrais vous dire quand même, ce sénateur que le meilleur moyen pour améliorer ma déjà dense, c'est qu'il y ait plus effectif et j'espère que vous voterez la recréation dès 11 unités de forces mobiles parce que quand vous avez plus. 2 policiers et de gendarmes spécialisés dans le public, vous les faites plus reposé et vous les faites plus formé parce que vous faites davantage les unités de forces mobiles quand vous en avez pas assez ben, vous les faites trop travaillé, je vous le disais tout à l'heure que je leur dois déjà cinq semaines de congés payés, ils sont fatigués, quand vous faites parfois, vous faites des centaines de de kilomètres dans des fourgonnettes qui ne sont pas très toujours reluisant tout loin de votre famille, lorsque vous avez pas du week-end pour vous reposer que vous êtes parfois insulter à longueur de manifestations, il arrive parfois que quelques manifestants puisse ne pas aimer la police nationale, ça peut exister, vous savez bien est parfois dans un climat de violence mais aussi de surveillance, parce que là pour le coup, les images, eux, ils les vivent et les villes sans contrôle de la CNIL, c'est le moins qu'on puisse dire, donc c'est vraiment parfois extrêmement difficile comme métier comme profession, vous passez des heures, des heures et des heures à être dans des moments de d'hyper violence vous sollicitez des policiers dont le le but n'est pas de faire de leur public mais de la sécurité publique, il y a les difficultés que nous connaissons, donc je veux dire que vous avez raison, vous n'avez pas évoqué les effectifs mais je veux vous dire que c'est une grande nouvelle pour la police de la République et leur public, de recréer ces escadrons de gendarmerie et ce serait que, malheureusement, plusieurs gouvernements ont ont supprimé en en 20 ans parce qu'on a supprimé 15 ans 20 ans pour qu'on puisse se reposer une partie de ces gendarmes de ces policiers et c'est le nombre qui fait le calme de la manifestation, quand vous avez beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes, les gens ne cherche pas la confrontation, quand vous avez moins d'effectifs, bah on voit qu'il y a des faiblesses dans le dispositif et ça peut créer soit la panique du côté des policiers, c'est tout à fait possible soit une envie d'en découdre pour ceux qui n'étaient pas venus comme des manifestants simplement autour d'une cause mais pour casser du flic, ça peut aussi arriver, donc je peux partager, je crois que je me range à l'avis du sénateur de Bresse, vous avez une mission, j'ai moi-même écrit un schéma c'est pas toutes tout à fait l'objet du texte aujourd'hui, mais c'est un débat extrêmement intéressant, j'espère surtout que vous voterez les augmentations d'effectifs et création du FN. Merci, alors je me vois l'amendement semaine de qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour, qui est contre. Qui s'abstient n'est pas adopté l'amendement 123 messieurs Merci madame la présidente, la commission des lois a fait le choix d'aborder la question du refus d'obtempérer, par un accroissement des sanctions dans l'article 7 bis du projet de loi. Je vais essayer de peser mes mots parce que c'est un sujet qui est extrêmement, extrêmement lourd, qui touche à des vies humaines la vie des policiers qui se trouvent parfois mis en danger par des refus d'obtempérer et la vie de ceux qui sont dans les véhicules, auteur de faits ou passager et j'évite ici la litanie des exemples récents de personnes qui ont été tués dans ces circonstances, fait aggravant, cette loi est une voix socialiste, donc je n'ignore pas et j'évite toute de suite les les arguments, c'est vous qui la votez oui, oui, il se trouve, il se trouve que des études récentes indiquent que, sans doute, la modification de la loi a induit plus de tirs policiers lors de refus d'obtempérer et que un certain nombre de vies humaines sont perdues à cause de cela, alors on a eu l'échange avec le ministre-dans un autre cadre, il est évident que la vie des policiers eux-mêmes et brisé dans ces circonstances, il est évident qu'il s'agit pour eux de se défendre, mais pour autant, on constate qu'il y a plus de tirs policiers mortel dans cette circonstance, alors que les autres tirs policiers sont moins mortel, on constate que même si il y a une augmentation des refus d'obtempérer, qui est manifeste, le nombre de personnes tuées les davantage encore dans des proportions plus importantes, c'est pourquoi nous proposons une modification de la loi qui n'est sans doute pas parfaite qui n'apportera pas toutes les solutions, mais nous sommes que ce sujet-là, il est vraiment central et on veut le dire avec beaucoup de gravité, beaucoup de solennité dans la qualité de la relation entre la police et la population et qu'il faut qu'on trouve une solution pour améliorer les choses de façon à ce que on ait plus cette actualité triste actualité de policiers qui tuent des contrevenants malheureusement. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur, je pense que c'est défavorable comme vous l'avez dit. Avis défavorable, on en est à en moyenne 75 refus d'obtempérer par jour. ça a augmenté de 28 % depuis 2015 le ministre lui-même a dit que quand malheureusement il accompagné les les personnes de leurs funérailles, c'était très souvent à cause de refus d'obtempérer et on voudrait désarmer les policiers dans ces conditions là, mais je pense que vous êtes complètement alors vous dites, il y a des études qui montrent que, oui, moi j'ai lu des études qui disent exactement le contraire : avis défavorable et j'aurai l'occasion de présenter un amendement qui va durcir fortement les sanctions contre les refus d'obtempérer, je pense que ce sera beaucoup plus efficace. Merci l'avis du gouvernement, même avis, merci, je me suis Durand. Vous remarquerez qu'on a plutôt dans ce débat tenu un certain niveau de dignité, de responsabilité, donc je j'entends les arguments de Marc-Philippe Daubresse que dont j'apprécie le travail, par ailleurs, personne, personne n'a parlé de désarmer les policiers. En revanche, dans une situation sociale qui est parfois tendu et il est possible qu'elle le soit dans les, dans les semaines à venir, ou dans les mois à venir davantage encore pour toute une série de raisons qui sont extérieurs à nos débats. Laisser prospérer des situations où on confronte la population aux policiers n'est pas responsable pour les parlementaires que nous sommes donc le sujet n'est pas de dire et en plus je l'ai dit tout à l'heure, c'est une loi socialiste, donc on pourrait être un peu discret sur le sujet, mais si on continue à avoir des faits de ce type, des passagers, des passants, des situations conflictuelles alors l'efficacité promise tout à l'heure par Marc-Philippe Daubresse, ça ne sera pas au rendez-vous, donc moi je veux bien qu'on se dise simplement on augmente le quantum de peine ont durci, ça suffit, Rabat ne ne nous nous pensons que ça ne suffira pas, ça ne suffira pas et il faut travailler autrement, le ministre a eu l'occasion de dire dans d'autres circonstances que il y avait pas d'armes intermédiaire entre finalement ne rien faire et tiré, il se trouve quand même que moi j'ai un peu confiance dans les travaux de fond qui sont conduits et quand on nous dit il y a sans doute dans le libellé de la loi des circonstances qui occasionnent ces pertes de contrôle cette difficulté de passer à l'acte quand parfois des commissaires à qui vous parlez, disent. Je reprends leurs mots, on a cette année de collègues qui ont utilisé leur arme hé ben moi, ça m'a posé un problème parce que je pense que c'était inadapté, voilà, je pense que notre responsabilité c'est de poser le la question au fond et c'est pas rester sur des solutions un peu facilement qui seront non mais j'ai même pas fini, madame qui seront inefficaces, excusez-moi, on va aller au bout. Monsieur le Ministre. Oui, j'ai j'ai pas pris la parole monsieur le monsieur le sénateur, parce qu'on aura un débat tout à l'heure, enfin tout demain ou après-demain sur l'amendement non déposé par le gouvernement, vous l'avez remarqué sur les refus d'obtempérer. c'est une question extrêmement difficile. Parce que personne ne peut satisfaire monsieur le sénateur. Du décès. Alors, évidemment, d'un policier ou un gendarme qui sont quand même eux aussi victimes, on l'a dit d'homicide, il y a pas d'autre mot. Ou de toute personne qui soit d'ailleurs contrevenante ou accompagnant le contrevenant. Qui viendrait à part de la vie dans un contrôle routier. évidemment, par nature, je vais évidemment le souligner. Personne ne peut non plus accepter que l'autorité de l'État soit à ce point bafoué que lorsqu'un policier, un gendarme dit Stop, on s'arrête pas. C'est aussi un peu embêtant pour l'autorité de l'État et vous êtes un républicain et évidemment si force doit rester à la loi, que faire devant tous les refus de tempérer tout et demi heure désormais toutes les demi-heures en zone police comme en zone gendarmerie. Peut-être que c'est une évidence qu'il faut rappeler, pardon de cette tautologie quand un policier, un gendarme s'approche, ce qu'on peut dire à nos concitoyens vous demande de vous arrêter, je propose que tout le monde s'arrête, ça me paraît ah béaba peut-être a rappelé et je sais que vous avez pas d'une averse, mais il y a pas de situation où tiens, il y aurait une égalité entre policiers et celui qui se serait pas arrêté évidemment, quelqu'un a commis un délit. Et très souvent on constate malheureusement, quelle que soit l'issue de ce refus d'obtempérer lorsqu'elle est la personne est arrêté, d'une manière ou d'une autre, soit il conduit sans permis et parfois ça s'aggrave soyez sous un état alcoolique ou un État stupéfiants, soit il a lui-même une recherché pour normalement de être en prison au lieu d'être dehors, soit il a de la drogue ou d'autres produits licites dans dans sa voiture, ils sont extrêmement rares, les gens qui, ayant un permis n'ayant pas consommé d'alcool de stupéfiants ne posant aucun problème à personne : tiens, se dit : je vais pas m'arrêter au contrôle de police, que, malheureusement, une grande partie des personnes qui sont arrêtés dans le cas de refus d'obtempérer ont par ailleurs en plus du délit qu'ils ont commis de ne pas s'arrêter. Quelque chose à se reprocher, comme on dit dans le langage policier, ça vaut évidemment pour nos amis douaniers qui vivent les mêmes choses, alors là il y a 3 sujets il y a un sujet statistique on est manifestement pas d'accord, mais peut-être que d'ici l'amendement proposé par le président Retailleau et rapporteur de Brest, on aura l'occasion d'en reparler j'ai déjà eu l'occasion de vous dire, monsieur le sénateur, mais je suis prêt à confronter bien sûr des parce qu'elles sont importantes qu'à ma connaissance. Il n'y a pas eu davantage de tirs. Par les policiers et par les gendarmes. Tout confondu. En 2021. Que en année 2016, 2017, c'est-à-dire avant la loi portée par votre majorité, il y avait même eu statistiquement moins si j'ai bonne mémoire, je n'ai pas trouvé ma fiche, en 2021 qu'en 2017, me semble-t-il, et même pendant les années Covid, où nous étions censés avoir moins de voitures qui circulaient en 2020, 2021, de mémoire, il y en a plus de 150 quand même, c'est-à-dire qu'il veut dire, refus d'obtempérer, même lorsqu'on avait pu conduire totalement sa voiture, ce qui prouve a bien souligné que ceux qui conduisent en voiture et qui font des refus de tempérer le fond y compris quand on leur interdise de conduire ce qui paraît d'ailleurs pas totalement illogique. Donc, il est faux, me semble-t-il, statistiquement, de dire que les policiers, les gendarmes tirent plus grâce ou à cause de la disposition des chétif que vous avez fait voter ou par manque de formation des policiers, des gendarmes, alors même que c'est sénateur de Brest a eu juste raison de rappeler qu'il y a eu plus, en moyenne, de refus d'obtempérer, il y a dans le cul, un peu moins de tirs statistiquement et plus de refus d'obtempérer, ce qui est vrai c'est qu'il y a eu plus de tirs mortels. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et la question qu'il faut se poser les donc triple. Est ce que les policiers gendarmes tirent plus et. La réponse est non, mais touche davantage les personnes qui soit conducteur ou accompagnant et entraîne leur mort est-ce que c'est le fait qu'ils ont une mauvaise formation dans le maniement de leurs armes, premières hypothèses. 2ème hypothèse, les personnes qui. Conduisent en voiture et font du refus d'obtempérer, prennent de plus en plus de risques. Et, désormais, ne se font pas simplement mine de pas s'arrêter mais fonce délibérément sur les policiers, les gendarmes.

de la voiture fonce vers le policier dans certains cadre déontologique, on peut sortir son arme et tiré, bon 3ème sujet. Nous avons une possibilité qui est celle de considérer que nous n'avons pas trouvé les moyens techniques qui consiste à à faire arrêter des véhicules par autre chose que par des armes à feu et c'est ce que je vous évoquais en disant que, à ma connaissance, mais moi je suis prêt à changer un certain nombre de choses, de même qu'on a inventé le LBD pour que les, les, les policiers et les gendarmes de tire pas armes à feu sur les manifestants, on peut toujours discuter de la capacité du LBD c'est quand même moins grave, moins létal car Revolver, bon c'est c'est c'est c'est fait, donc on a inventé une arme intermédiaire dans des manifestations, on peut toujours discuter évidemment de de une saison de cette arme, ce que vous voyez ce que je veux dire la démonstration donc là aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, que je suis n'a pas d'arme intermédiaire pour faire arrêter un véhicule entre l'arme à feu rien. La loi sécurité globale a avancé puisqu'nous a permis, on en a parlé de maître des sticks sans autorisation judiciaire parce que jusqu'à présent n'y compris les polices municipales ne pouvait pas utiliser les sticks, sans qu'on soit, officier de police judiciaire, c'est absurde, mais c'est comme ça. Donc quelques sénateurs de Brest, nous l'avons fait entre guillemets sauter dans le texte de loi mais ça suffit pas, bien évidemment, donc je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus, me semble-t-il, un peu moins définitif sur pourquoi il y a davantage d'accidents mortels ou de tentative d'homicide, ça dépend comment on regarde les choses, alors je terminerai par dire, Monsieur le Sénateur que. C'est toujours un débat très difficile parce que dans une soirée sénatoriales comme celle-ci où dans la. Moteur et le confort de mon bureau et vous évoquez des commissaires de police, j'ai beaucoup de respect pour commissaire de police, mais je trouve que c'est rarement, eux qui sont à deux heures du matin avec le policier a joint sur une route de du Lot-et-Garonne, mais ce que je veux dire, donc je j'ai beaucoup de respect pour les commissaires de police, mais

mais je me mets aussi 20 secondes à la place, quand je vais voir les effectifs ou quand je les appelle des 2 types qui vous disent : écoutez, monsieur le ministre, il était 3 heures du matin, il faisait nuit, ça fait 5 ans qu'on était dehors, il faisait froid, il y avait pas de lumière, il y a déjà trois mecs qui ont fait, refus d'obtempérer, juste avant, et la France sont mon collègue

tous études sociologiques tous tes études sur la formation, il faut sans doute les faire c'est pas une nature faut pas penser à la fin des fins, c'est pas nous qui sommes devant ces véhicules qui font ça vite à 100 à 100 50 kilomètres à l'heure où les pères et mères de famille que sont les policiers, gendarmes, se disent qu'est-ce que je fais, il y a sans doute des moments où on peut se dire peut-être que c'est excessif. Ben de toute façon, quoi qu'il arrive sa justice en décider il y a ceux des moments où on se dit on peut comprendre le comportement d'ailleurs, je constate que, souvent, lorsque les médias font un zoom sur une affaire assez vite, on ne parle plus de l'affaire et dans les jours après, alors qu'il serait intéressant, avec un peu de calme, de regarder où ça en est. Voilà par exemple une belle action de l'IGPN j'ai peiné gégène met systématiquement en garde à vue, les policiers qui ont tiré, même s'ils sont parfaitement dans leur raison et attends à certains nombres de décisions de justice du procureur de la République pour savoir s'ils ne sont pas poursuivis et beaucoup de policiers, sont mis en examen en attendant une décision plénière, si j'ose dire, du juge siège si j'ose dire, non pas par précaution mais pour montrer que, on ne laisse pas faire de la pente quoi, des gens qui portent la violence légitime, donc on peut pas dire non plus parce que le sénateur mais vous savez bien que quand un policier tire, il se passe rien derrière, pour lui, c'est toujours un problème personnel juridique. et, bien sûr, humains, voilà donc moi je trouve que cette question est très importante, je ne voudrais pas puisque vous prenez la parole pour dire il faut sans doute davantage encadrée, je l'entends bien qu'on se dise que ce soit une discussion qui ne prend pas en compte non plus la grande détresse de l'autorité de l'État, lorsqu'un policier, un gendarme dit Stop et qu'on ne s'arrête pas, et je pense que, quels que soient ceux qui sont au pouvoir, c'est une question qui se pose. Merci, alors je vais mettre voit donc l'amendement 123 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient n'est pas vous adoptez alors Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il est maintenant un peu plus de minuit, je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à minuit et demie afin d'aller plus avant dans l'examen de ce texte, enfin un petit peu plus avant,

Le comité d'éthique prévues par le rapport annexé relève d'une excellente idée, évaluer l'action du ministère de l'intérieur par une instance spécialisée. Nous trouvons que ça va dans le bon sens mais, comme souvent, et comme dans d'autres parties du rapport la rédaction actuelle ne permet pas d'avoir les garanties nécessaires pour un fonctionnement efficace, il est écrit que ce comité sera placée auprès du ministère de l'Intérieur, nous souhaitons au contraire mon mentionné qu'ils seraient indépendants, nous souhaitons également qu'il soit présidé par le défenseur des droits, dont les missions ne sommes parfaitement en adéquation avec les attendus du comité, ce qui permettra d'avoir des garanties nécessaires sur son indépendance, il est écrit que ce comité sera composé de personnalités qualifiées indiscutable alors nous trouvons que cette rédaction est tel particulièrement discutable et qui allaient plutôt vide de sens, c'est pourquoi nous proposons qu'il soit composée de représentants du monde universitaire, chercheur en criminologie en sociologie et dans toutes les branches essence humaine et sociale, intéressé par les questions de sécurité, mais aussi des représentants du monde associatif et de la population afin d'avoir une véritable représentation au service de l'efficacité du comité nous souhaitons également lui ajouter quelques sujets parmi les exemples de thématiques qu'il pourrait avoir à traiter comme le maintien de l'ordre ou les relations police-population, nous souhaitons aussi que les recommandations émises par ce comité soient rapidement prises en compte par le ministère, rien ne serait plus inutile que de transformer ce comité en usine à produire des rapports que personne ne lit ou ne met en oeuvre, ensuite, nous souhaitons que l'action du comité d'éthique, fasse l'objet d'un compte-rendu annuel au Parlement afin de nous permettre dans l'hémicycle et en commission de nourrir davantage nos réflexions sur le contrôle de l'action du gouvernement en matière de sécurité et véritables, comité d'éthique efficace et indépendant, voilà notre ambition.

je pense que sur ce point, nous sommes tous d'accord, tout citoyen libres de manifester pacifiquement, sans avoir à que Red Hat fichier fouillé, identifié par les autorités publiques, or cette pratique est aujourd'hui limité à les limiter, d'abord par les violences au sein des cortèges bien entendu et elle est limitée aussi par un recours quelquefois disproportionnée à l'usage de la force et des armes par les forces de l'ordre ces tensions décourage les personnes vulnérables accompagné d'enfants par exemple ou âgé de participer à des manifestations. Il est temps de mettre en oeuvre, nous semble-t-il, une autre doctrine du Mathias de l'Ordre qui permettrait à la fois un recours à la force plus proportionnée et également de choisir une approche destinée à pacifier les rapports et à sortir d'une logique de confrontation permanente. Le groupe Écologie solidarité et territoires appelle de ses voeux l'interdiction de la pratique des NAS consistant serrer les manifestants à l'intérieur de cordon policier cette pratique représente un réel danger en cas de mouvement de foule, il appelle également à encadrer l'usage de grenades lacrymogènes lors des manifestations, une utilisation abusive de ces grenades pouvant générer de grandes tensions, mouvement de foule et blessures comme cela a été constatée et démontrée par la commission du Sénat lors des incidents au Stade de France le 28 mai 2022 à Saint-Denis. Merci l'avis de la commission sur ces deux amendements. Tous les amendements relatifs à l'IGPN au maintien de l'ordre pour les raisons que j'ai exposées précédemment défavorable. Merci même avis merci donc je mets aux voix l'amendement 146. Qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour,

Roche. Découle d'une proposition de la Cncdh dans son avis du 11 février 2021 sur les rapports entre la police et la population concernant les enquêtes administratives, la commission s'est interrogé sur la pertinence, en termes de compréhension et de lisibilité du système de l'existence d'une pluralité d'acteurs susceptibles de recevoir un signalement. Le groupe Écologie solidarité et territoires demande donc au gouvernement de mettre en place une plateforme unique de signalement des manquements à la déontologie commune aux défenseurs des droits à l'IGPN et à l'hygiène. défavorable merci je mets aux voix, donc oui monsieur Ménard Roche. Non, simplement je remarque que les avis sont de plus en plus bref donc défavorable, j'ai toujours pas compris mais enfin peu importe pourquoi, en fait, je voulais juste il est tard, certes, mais enfin, on est là pour un certain temps encore demain, après-demain, il me reste une minute 47 donc, en fait, il était, mais le sujet est grave, je, je dis juste que je remarque que les repas sont de plus en plus brève et j'aimerais bien avoir des arguments certaines fois qu'il m'explique pourquoi c'est pas bon, à part le rapport bien entendu monsieur Dobres que nous attendons bien entendu, ça je comprends. Merci. Ce qui a une mission d'information qui est lancé et que franchement à chaque fois refaire des amendements qui préjuge de ce que cette mission peut donner comme proposition ou énoncé comme garantie s'est cassé le travail des collègues qui sont d'ailleurs pluraliste dans cette mission, voilà ce que je dis, et voilà pourquoi nos avis sont défavorables. Merci, alors je mets aux voix l'amendement dans 83. Il a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient n'est donc pas adopté l'amendement 200 Mais la présidente assassine. Oui merci madame la présidente, je veux simplement dire à monsieur le rapporteur, que nous ne faisons qu'user de notre droit d'amendement. donc effectivement il y a peut-être des choses redondantes ou des missions qui sont en cours mais rien ne nous empêche de déposer des amendements pour éclaircir ou peut-être avancer aussi sur un certain nombre de questions qui qui qui viendront, mais c'est notre droit d'amendement, mon cher collègue, les constitutionnelle, je vous le rappelle, donc, sur cet amendement 200 hein, nous souhaitons garantir l'effectivité du suivi des plaintes à l'IGPN aujourd'hui, si une personne pense être victime ou témoin d'un comportement illégal d'un agent de la police nationale, elle peut saisir en ligne, l'inspection générale de la police nationale IGPN la victime de ce comportement utilise alors un formulaire de signalement en ligne, mais ce n'est que si elle le souhaite, qu'elle sera informé des suites données à celui-ci, l'information est donc facultative en revanche la plateforme précise que toute dénonciation mensongère et systématiquement signalé à l'autorité judiciaire et peut faire l'objet d'une plainte du ministère de l'Intérieur, on passe donc du signalement à l'issue incertaine pour la victime d'un comportement illégal d'un agent de police à une dénonciation systématique en cas de potentiel dénonciation mon mensongère, c'est pourquoi nous souhaitons garantir l'effectivité du suivi des plaintes à l'IGPN et de leur traitement en instaurant un délai de traitement des plaintes par l'IGPN deux 3 mois sur le modèle de la plainte judiciaire avec une obligation de suivi. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur défavorable, merci la vie de gouvernement Monsieur le Ministre.

je ne peux pas donner un avis favorable par principe parce que je sais pas si trois mois sont sont possibles, mais je peux m'engager vis-à-vis de vous pour vous adresser, je regarde mon cabinet peut être la moyenne avec laquelle on traite ces difficultés là et peut être m'engager à donner d'instructions pour que si jamais c'est trop long, je j'en sais rien, j'ai essayé d'avoir les chiffres de c'est pas eu ces derniers jours, parce que je crois que l'une des difficultés que nous avons c'est que il souvent les personnes qui, sur la plateforme de signalement signale des choses ne signale pas tout d'un seul coup, et qu'il faut faire un certain nombre d'enquêtes pour savoir si ce policier, par exemple, il existe, il travaille bien, ce jour là, ces personnes, de bien donner davantage d'éléments avait-il ces caméras-piétons et donc, vous voyez une phase d'instruction qui empêche parfois de donner les statistiques, de statistiques de globales, je voudrais quand même souligner que lorsque le président de la République avait évoqué sa plateforme contre les discriminations. Beaucoup ont cru que ce serait la police nationale ou la gendarmerie nationale qui arriveraient les premiers, sachez que nous étions la dernière administration qui avait été évoqué ce discrimination je crois de mémoire, monsieur le rapporteur de ce que les questions autour du logement, les questions autour de la santé, les questions autour d'un axe certain nombre d'accès au service public était bien devant nous dans les signalements faits sur la discrimination que les services de police et gendarmerie de mémoire, on devait être autour de 7 % de l'ensemble de signalements c'est 7 % de trop, je ne le nie pas, mais ce que je voulais dire c'est que, contrairement à l'idée répandue que ce serait les policiers gendarmes qui ferait le plus de discrimination, c'est le logement en 1er et puis l'accès à l'emploi, mais vous connaissez c'est ce sujet mieux que moi, je terminerai pas dire que c'est là où je me dis que je ai mon mes devoirs et j'aurais dû publier le rapport de monsieur Chantepy, que vous connaissez bien, qui, non c'est pas ce c'est pas c'est pas monsieur, qui est du Conseil d'État, je, je commence à être fatigué, monsieur Vigouroux, voilà, c'est un conseil d'État mais honorable mais et respectueux et respectable, pardon, mais je, je les avais confondu, qui a fait un important rapport que je lui ai commandé voilà plusieurs mois désormais très intéressant qui qui évoque la discrimination dans les forces de sécurité intérieure et il évoque 3 types de discrimination des premières ces dissimulations dont l'auteur sont les forces de sécurité intérieure. Personne ne dit le contraire, une situation qui ne sont pas simplement des discriminations qui peut être fondée sur le nom ce faciès, ça peut être sur l'orientation sexuelle, par exemple, le bien évidemment, mais les des discriminations autour du genre du sexe, voilà donc il est très documenté

Il y a aussi dans des services de police dans des services de gendarmerie, des personnes qui subissent les discriminations parce que ce sont des femmes, parce que ce sont des homosexuels parce que ils viennent de telle ou telle origine géographique et que nous ne pouvons pas moi en tant qu'employeur ignorer ce fait, elles sont certes pas importante, mais elles existent et, parfois, elles font naître ici des suicides, là, des difficultés de quitte uniforme et cetera et je me sens responsable une partie de ses distributions, bien évidemment 3ème ce que j'évoquais tout à l'heure. Discrimination, c'est ce que subissent ces forces de l'ordre. Et je l'ai dit de subissent aussi quand c'est des femmes qui contrôle en certains endroits un peu difficile, elles ont des difficultés de sa respecter non pas l'uniforme qu'elle porte mais le genre qu'elles sont.

ou de gens qui sont de couleur de peau différente et donc je pense que quand on regarde les discriminations je je ne sais pas ce que vous avez dit la la sénatrice mais je dis pour tout le monde, il faut regarder le fait qu'ils sont aussi responsables de ces, de ces discriminations donc ce que je propose, monsieur le président de la commission des lois, c'est que je je rendrai public ce rapport, je vous laisserai peut-être de faire communiquer l'ensemble des membres de votre commission et peut-être de du Sénat, il est extrêmement instructif et nous suivrons ces recommandations. Merci, alors je mets aux voix donc l'amendement 200 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour,

parce que Monsieur Durand a eu l'occasion de défendre le sujet qui qui est inscrit dans cet amendement, donc je ne serai pas redondantes et quant aux 200 en fait, c'est une erreur de notre part et je le regrette puisqu'effectivement il y a déjà une magistrate qui a été nommé à la tête de l'IGPN merci

ayant dénoncé des actes de racismes et de maltraitance qu'on met régulièrement par des agents de police dans les cellules du dépôt du tribunal judiciaire de Paris a été sanctionné pour avoir témoigné de son vécu à l'Assemblée nationale son engagement à faire cesser ces faits de racisme et maltraitance a débuté par un signalement en interne, puis par un signalement aux autorités compétentes, dont l'IGPN sans retour des autorités et après plusieurs pressions qu'il subissait en interne, monsieur ben Mohamed a dévoilé les faits dans les médias son combat ainsi que celui d'autres lanceurs d'alerte dans la gendarmerie dans la police relève pourtant de l'intérêt général, il en va de la dignité de nos concitoyens et de la confiance entre les forces de l'ordre et de la population, les agents de police et de la gendarmerie sont soumis comme tout fonctionnaire, devoir de réserve, mais ils sont souvent confrontés à une absence de réactions de leur hiérarchie lorsqu'ils transmettent des informations et des dysfonctionnements internes, exposés à des risques de pressions et des menaces, ils sont dissuadés de dénoncer les faits dont ils sont témoins. Certains agents se trouve prisonnier de l'Arctique 40 qui le leur permettrait que signalement judiciaire tout ceci rend étrange tout positionnement qui voudrait que l'article 40 du code pénal protège du déclarant pour ces raisons, le groupe écologiste solidarité et territoires demande à ce que la protection du statut de lanceur d'alerte, telle qu'elle réside, de la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte soient accordée aux agents des forces de l'ordre. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. La loi du 21 mars 2022 sur les lanceurs d'alerte, a fait l'objet d'un large débat ici a été tranchée par notre commission et ensuite par les assemblées parlementaires et par ailleurs, l'article 40 du code de procédure pénale est très clair et les et donc la demande de monsieur Ménard Roche est satisfaite de fête : avis défavorable. Merci même avis merci donc je vais mettre aux voix l'amendement 84 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient n'est pas adopté, mes chers collègues. Je vais lever la séance, nous avons examiné 66 amendements sur ce texte, il en reste 138 à examiner prochaine séance mercredi 12 octobre à 15 heures pour les questions d'actualité au gouvernement et la séance est levée.